La séance est reprise. L'ordre du jour appelle les explications de vote sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à lutter contre le mitage des espaces forestiers en Île-de-France (proposition n° 159, texte de la commission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

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les problématiques urbaines, très prégnantes en Île-de-France, ne doivent pas occulter les enjeux agricoles et forestiers qui se concentrent aussi dans cette région, en particulier dans la grande couronne

Malgré la bonne volonté des collectivités locales et l'action de l'Office national des forêts, certaines zones forestières se dégradent pourtant. Lequel d'entre nous n'a-t-il pas déploré des dépôts sauvages en lisière de forêt ? On recense aussi, un peu partout, des surfaces en déshérence bloquées par l'indivision. autre fléau a reçu le nom de « cabanisation » : il s'agit des constructions illégales qui affectent les zones naturelles. Enfin se pose la question du mitage, qui nous intéresse directement aujourd'hui.

qui entraîne une pression foncière très conséquente. Le mécanisme est bien connu : certains propriétaires profitent de cette pression pour vendre de petites parcelles à des prix très élevés, dans la perspective de leur changement d'affectation. Ces pratiques destinées à la réalisation d'opérations juteuses sont l'un des obstacles à la bonne gestion de nos forêts. Elles accentuent un morcellement déjà très ancré sur notre territoire du fait de l'existence ancestrale d'une multitude de propriétaires privés. privés. Bien des outils spécifiques à la région francilienne peuvent être mobilisés pour protéger les espaces naturels, notamment l'agence des espaces verts de la région, ou encore les conventions de surveillance et d'interventions foncières qui réunissent la Safer et les collectivités locales. ces leviers ne suffisent pas à prévenir radicalement le mitage des espaces forestiers. Aussi, je salue l'initiative de nos collègues députés visant à reconduire le dispositif expérimental adopté dans le cadre de la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain. Il s'agit- cela a été rappelé -de pérenniser le droit de préemption de la Safer l'Île-de-France pour les espaces boisés d'une superficie inférieure à trois hectares. Le bilan de l'expérimentation réalisée depuis plus par la Safer semble démontrer son efficacité, puisque 198 préemptions sur 510 ont été effectuées au titre de la protection et de la mise en valeur de la forêt. La taille des parcelles concernées, qui s'établit en moyenne autour de 5 000 carrés, répond à l'objectif précis de lutte contre le mitage. Bien entendu, malgré la qualité des missions exercées par la Safer d'Île-de-France, cet outil préventif ne résoudra pas tout. Lutter contre la spirale du mitage impose une vigilance à bien des égards. peut notamment passer par une mise à jour rigoureuse des parcelles forestières en déshérence, par l'application efficiente des sanctions prévues à l'encontre des bâtis illégaux, ou encore par l'appel au respect des règles déontologiques par les acteurs impliqués dans les ventes de petites parcelles forestières.

qui prévaut sur ce texte. Mes collègues et moi-même y sommes d'autant plus favorables que l'objectif de lutte contre le mitage et, plus globalement, contre le morcellement contribue à répondre à un autre défi, celui de la sous-exploitation de la forêt française en général.

en dépit de nombreux dispositifs publics de soutien, la structuration de la filière bois n'est pas encore optimale, ce qui est bien regrettable. Cela dit, je tiens à répéter que la forêt est un bien commun que l'urgence écologique nous impose de conserver. L'accord de Paris sur le climat le rappelle, à son article 5, en invitant à l'instauration de mesures contre le déboisement. En adoptant ce texte, nous apporterons ainsi une petite contribution à l'effort collectif de protection des zones naturelles.

nous n'avons pu que constater la violence inédite des incendies meurtriers qui dévastent l'Australie, sa faune et sa flore. Si la préservation du patrimoine forestier mondial prend, à l'aune du changement climatique, une importance particulière, l'inquiétude quant à l'état des forêts françaises est ancienne. En effet, notre forêt tempérée associe des organismes vivants, végétaux et animaux, de toutes sortes et de toutes tailles, à des milieux très diversifiés par les sols, les climats, l'eau et les matières minérales. Comme tout être vivant, notre forêt est soumise à des influences susceptibles de perturber un équilibre fragile. Mitage forestier, phénomène de « cabanisation », pollution : les menaces sur la forêt française, si elles ont changé de visage, demeurent d'actualité. L'action indispensable du garde forestier ne suffit plus. La préservation de la forêt requiert l'intervention du législateur. de loi que nous examinons aujourd'hui a été déposée par le député Jean-Noël Barrot, vise à lutter contre le mitage des espaces forestiers en Île-de-France. Pour rappel, le mitage n'est autre que la vente de parcelles de petite taille à des particuliers, souvent à des prix très élevés, en vue de donner au bien ainsi acquis un usage non conforme à sa vocation naturelle ou à son classement dans les documents d'urbanisme locaux. L'île de France est, malgré son caractère urbain remarquable, aussi verte que bien d'autres régions françaises : ses 261 000 hectares de forêts aux caractéristiques bien spécifiques justifient la mise en oeuvre d'outils spécifiques concourant à la préservation de cette forêt. En effet, le poumon vert de la région la plus densément peuplée du pays est soumis à une pression foncière sans comparaison avec le reste du territoire

La forêt francilienne apparaît donc, dans ce contexte, particulièrement exposée au mitage forestier. L'objectif de cette proposition de loi est simple : il s'agit de pérenniser un dispositif expérimental.

d'une superficie totale inférieure à trois hectares, lorsque l'exercice de ce droit de préemption a pour objet la protection et la mise en valeur de la forêt desdites parcelles. L'expérimentation n'est pas encore arrivée à son terme.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : depuis février 2017, la Safer d'Île-de-France a engagé de la sorte 198 préemptions. Ces actions ont été fréquemment motivées par plusieurs objectifs légaux, mais, dans 107 cas, le principal objectif invoqué était la protection et la mise en valeur de la forêt. En d'autres termes, si nous n'avions pas légiféré sur le sujet et mis en place cette expérimentation il y a trois ans, dans 107 cas, soit 20 % des situations de préemption, les collectivités et la Safer se seraient trouvées impuissantes face à une vente contribuant à accroître le mitage L'efficacité de ce dispositif sur le territoire repose sur son caractère préventif. C'est bien logique, puisque, une fois la parcelle vendue, illégalement défrichée et artificialisée, il est particulièrement difficile pour les communes d'intervenir. Je le redis : des collectivités territoriales à la Safer, des propriétaires privés aux préfectures, en passant par les associations environnementales, tous les acteurs sont d'accord quant à la qualité de ce dispositif, qui a fait la preuve de sa pertinence opérationnelle. Mes chers collègues, les objectifs fixés dans le cadre de l'expérimentation- amélioration de la structure des propriétés forestières et préservation des forêts franciliennes du mitage, de la pression foncière et de l'étalement urbain -ayant été atteints,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, votée le 28 novembre dernier par l'Assemblée nationale, la proposition de loi visant à lutter contre le mitage des espaces forestiers franciliens a été adoptée, suivant la procédure de législation en commission, par la commission des affaires économiques.

En effet, nous pensons qu'il faut aborder cette proposition de loi dans le contexte plus global de l'urgence écologique et de l'impérative nécessité de protéger notre patrimoine forestier. Comme le souligne l'accord de Paris sur le climat, les forêts et les arbres jouent un rôle essentiel, agissant comme des puits de carbone et absorbant l'équivalent de 2 milliards de tonnes de dioxyde de carbone chaque année. Or la forêt française est la troisième forêt d'Europe : elle occupe 30 % du territoire national et capte chaque année près de 70 millions de tonnes de CO2. Avec près de 140 variétés d'arbres différentes, elle compte parmi les plus diversifiées d'Europe.

En Île-de-France, puisque tel est le champ géographique de la proposition de loi, la forêt est présente sur environ 261 000 hectares, soit un taux de boisement de 21 %, pour une moyenne nationale de près de 30 %. Or l'une des caractéristiques de cette surface forestière et boisée est son extrême morcellement, trois fois supérieur à l'échelle nationale, mais également son manque d'entretien. manque d'entretien. Comme cela a été souligné lors des travaux de la commission, cette situation accélère sa dégradation et favorise la spéculation. Le mitage forestier, la « cabanisation », l'artificialisation des sols, la pollution la dépose illégale de déchets, accélèrent la vente de parcelles de petite taille à des particuliers, à des entreprises ou à des fonds d'investissement, souvent à des prix très élevés. C'est pourquoi la proposition d'inscrire de manière pérenne dans la loi un droit de préemption à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Île-de-France pour les ventes de parcelles forestières de moins de trois hectares, lorsque l'opération vise à protéger et à mettre en valeur la forêt, est plus que nécessaire, d'autant que les collectivités se trouvent démunies pour freiner ce phénomène de mitage et de détournement de la fonction première de ces parcelles. En effet, depuis 2017, la Safer de l'Île-de-France a motivé, notamment par l'objectif de protection et de mise en valeur de la forêt, 198 préemptions. Ces actions ont été fréquemment justifiées par plusieurs objectifs légaux, mais, dans 107 cas, le principal objectif invoqué était la protection et la mise en valeur de la forêt. Ainsi, en l'absence de cette disposition, dans ces 107 cas, soit environ 20 % des préemptions de la Safer, celle-ci n'aurait pas pu empêcher la vente des parcelles et l'accroissement du mitage forestier qui en aurait résulté. Les 198 ventes sur lesquelles la Safer est intervenue représentent une surface totale d'environ 105 hectares de foncier forestier. Enfin, nous tenons à rappeler que, depuis de nombreuses années, notre groupe porte des amendements visant à élargir le droit de préférence des riverains, mais aussi à étendre, sur l'ensemble du territoire, le droit de préemption des Safer, ainsi que des communes forestières, aux parcelles boisées de moins de 4 hectares, ou encore à modifier le mode de représentation des Safer, en augmentant le nombre d'élus locaux et de la société civile. La forêt est devenue une valeur refuge, qui suscite beaucoup d'appétit de la part des investisseurs privés, lesquels n'ont que peu de considération pour l'écosystème forestier, pourtant si fragile. Et c'est encore plus prégnant en Île-de-France. C'est pourquoi, je le répète, nous voterons avec plaisir cette proposition de loi. La parole

revêt un caractère tout particulier, alors que plus de 10 millions d'hectares ont été détruits en Australie par de violents incendies depuis septembre dernier, laissant des paysages lunaires et des forêts dévastées. Les forêts constituent l'un de nos atouts majeurs dans la lutte contre le dérèglement climatique. Elles absorbent en effet chaque année 2 milliards de tonnes de CO2, l'un des principaux gaz à effet de serre. La France a la chance d'avoir 30 % de son territoire couvert par la forêt, ce qui lui permet d'absorber 70 millions de tonnes de CO2 chaque année. Les espaces forestiers sont également indispensables à la préservation de la biodiversité des espèces animales et végétales. Ils présentent des qualités environnementales évidentes, mais aussi des qualités sociales, comme point de contact entre l'homme moderne et la nature, et des qualités économiques, au travers de la sylviculture. Les forêts subissent cependant de nombreuses atteintes, et leur surface a continué, au cours des trente dernières années, à se réduire à l'échelon mondial. Parmi ces atteintes, les activités humaines jouent un rôle majeur, que ce soit pour la création d'espaces agricoles ou pour l'exploitation industrielle. Les feux de forêt, comme les incendies spectaculaires en Australie ou dans la forêt amazonienne, rendent la déforestation bien visible. Celle-ci révolte à juste titre les citoyens soucieux de l'environnement. Il existe cependant des menaces plus silencieuses et moins visibles. Le mitage en fait partie. Cette pratique, qui consiste en la vente de petites parcelles forestières à des particuliers, pour des usages qui ne correspondent pas à la destination de ces lieux, met en péril la croissance de nos forêts. La région de l'Île-de-France concentre un cinquième de la population française sur moins de 3 % de la superficie nationale. Malgré cette forte densité, la région parisienne comprend d'importantes surfaces boisées, représentant 20 % de son territoire. Élue de la Seine-et-Marne- le plus vaste département de l'Île-de-France -, où la forêt représente 25 % de la surface, vous comprendrez que je suis sensibilisée à ce sujet, d'autant que mon département reste le premier de la région pour la production de bois. Je ne puis non plus passer sous silence le massif de Fontainebleau, seconde forêt domaniale de France, qui s'étend sur 25 000 hectares. Pour tenter de protéger ces espaces contre le mitage, une expérimentation a été introduite par la loi de 2007 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain. Il s'agissait de conférer à la Safer Île-de-France un droit expérimental de préemption portant sur les parcelles forestières de moins de trois hectares. Le droit de préemption permet une intervention en amont, avant que la parcelle ne perde ses qualités forestières. Un tel dispositif permet d'entraver au minimum la liberté des propriétaires, qui demeurent maîtres de la décision de vendre leur parcelle et d'en fixer le prix. Cette expérimentation s'est révélée utile. Le bilan fait état de près de 200 préemptions, pour une surface moyenne de 5 000 mètres carrés par vente. Les différents acteurs de ces ventes ne se sont pas montrés hostiles au dispositif. Les collectivités locales sont à l'origine de la majorité des préemptions et, même si elles sont moins nombreuses, certaines préemptions ont eu lieu sur l'initiative de propriétaires privés. de loi que nous examinons aujourd'hui vise à rendre permanent le droit de préemption de la Safer Île-de-France. Ce texte peut sembler modeste, technique, mais nous pensons qu'il contribue utilement à la préservation de la forêt francilienne. Une question pourrait se poser quant à l'opportunité d'étendre ce dispositif à tout le territoire national, ou encore de le limiter aux zones soumises à une pression démographique ou à un étalement urbain important. Les résultats de l'expérimentation ont démontré l'efficacité et la pertinence du dispositif sur le territoire francilien, mais ces résultats ne valent que pour ce territoire, si particulier, avec ses 1 014 habitants au kilomètre carré. Le groupe Les Indépendants estime que toute atteinte à la liberté doit être strictement limitée et proportionnée au regard de l'objectif visé. L'éventuelle extension du mécanisme devra donc être soumise à un examen précis des spécificités de chaque territoire. Concernant la région d'Île-de-France, à l'heure où les enjeux climatiques et environnementaux sont devenus primordiaux, et dans un contexte régional où 98,8 % du territoire correspond à une aire urbaine, chaque hectare compte. Nous soutenons donc cette proposition de loi, qui, au vu de l'expérimentation, constitue une réponse adaptée au mitage des forêts franciliennes. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la forêt française constitue un des atouts naturels majeurs de la France, singulièrement dans le contexte actuel de transition énergétique et écologique, de lutte contre les gaz à effets de serre. Filière économique de tout premier plan, elle représente plus de 440 000 emplois répartis sur l'ensemble du territoire. Son potentiel de développement est considérable et nous ne sommes qu'aux prémices de ce que ce matériau renouvelable de substitution peut nous offrir. Cette forêt est aujourd'hui menacée, comme la plupart des espaces naturels. Victime de multiples fléaux, dont l'accélération du changement climatique n'est pas le moindre, elle pâtit aussi de l'étalement urbain. Ainsi en Île-de-France, elle est victime d'une urbanisation « sauvage » et d'une pression foncière toujours grandissante. Le mitage et la « cabanisation », tels qu'ils vous ont été expliqués, conduisent au « grignotage » et à la disparition de forêts périurbaines, pourtant plus que jamais essentielles à l'équilibre des régions densifiées. Ces constructions illégales font fi de l'autorité des maires et de leurs projets d'aménagements. Elles causent des nuisances aux riverains, entraînent des coûts supplémentaires à la charge directe et indirecte des collectivités, conduisent parfois à des extensions inopportunes de réseaux et rendent plus difficile la prévention des risques d'inondation, d'incendie et d'écoulement de boue. La principale mesure de ce texte consiste donc à pérenniser le dispositif de lutte contre le mitage forestier en Île-de-France, expérimenté depuis 2017. Il devenait urgent d'agir en mobilisant les outils existants, mais surtout en renouvelant l'action publique en la matière. En trois ans, le droit de préemption de la Safer Île-de-France a été utilisé 190 fois environ, souvent à la demande des collectivités locales. Cette proposition de loi est plébiscitée, tant par les élus locaux que par les forestiers. Le groupe centriste la soutiendra donc, tout en demandant que l'évaluation de ce droit de préemption, prévue dans la loi de 2017 à l'issue de l'expérimentation, puisse bien faire, monsieur le ministre, l'objet d'un débat, de manière à définir s'il est ou non pertinent de le dupliquer à d'autres espaces naturels périurbains. En effet, si la pression foncière et démographique est particulièrement forte en Île-de-France, elle s'accroît également aux abords d'autres métropoles. Face aux enjeux de climat, de neutralité carbone et de pollution, dans le cadre des PCAET, la place et les services rendus par les espaces forestiers sont devenus des sujets incontournables, qu'il convient de maîtriser, notamment tant que la fiscalité sur le foncier restera défavorable aux espaces naturels. Tant qu'il sera fiscalement plus intéressant d'urbaniser une parcelle que de préserver des espaces naturels, la tentation sera grande, et la disparition des espaces naturels risque de se poursuivre. Ce dispositif, utile pour lutter contre le mitage des espaces forestiers en Île-de-France, s'accompagne fort heureusement sur ces territoires périurbains, et depuis la mise en place des plans régionaux forêt-bois, de politiques de préservation et de développement forestier.

L'enjeu est tout autre, puisqu'il s'agit non pas d'éviter la « cabanisation », objet de ce texte, mais bien, pour lutter contre le morcellement, de permettre des regroupements de parcelles propices à créer des unités de gestion sylvicole durable.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la pédagogie étant affaire de répétition, je rappelle pour la énième fois que la proposition de loi n° 159, adoptée par l'Assemblée nationale et visant à lutter contre le mitage des espaces des espaces forestiers en Île-de-France, a pour objectif de pérenniser une expérimentation lancée il y a bientôt trois ans. Ce dispositif expérimental a démontré son utilité sur le terrain, mais il arrive bientôt à son terme et risque de s'éteindre si nous n'intervenons pas pour le pérenniser. Il s'agit donc de protéger la forêt francilienne. Ce « poumon vert » de la région la plus densément peuplée de l'Hexagone est en effet particulièrement exposé au phénomène de « mitage forestier Concrètement, des parcelles de petite taille sont vendues à des particuliers pour un prix élevé et font ensuite l'objet d'un usage non conforme à leur vocation naturelle ou à leur classement dans les documents d'urbanisme. Il en résulte un processus de « cabanisation Le mécanisme retenu pour contrecarrer cette évolution a été de créer un droit de préemption des petites parcelles forestières, au profit de la seule société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Île-de-France. Le succès de l'expérimentation est le critère fondamental pour permettre au législateur d'évaluer le bien-fondé d'une pérennisation. C'est également une condition de validité essentielle selon le juge constitutionnel celui-ci vérifie en effet que la pérennisation ou la généralisation d'un dispositif dérogatoire repose bien sur une évaluation de sa mise en oeuvre solide et convaincante. Or le bilan de la mise en oeuvre du nouveau droit de préemption du 28 février 2017 au 31 octobre 2019, transmis par la Safer Île-de-France, montre bien la nécessité de pérenniser le dispositif. En effet, sur presque 200 cas de mise en oeuvre du droit de préemption de parcelles forestières, la moitié n'aurait pas été possible sans actionner le dispositif expérimental. Plus en détail, quantitativement, depuis février 2017, l'objectif de protection et de mise en valeur de la forêt a figuré parmi les motifs invoqués par la Safer dans 198 procédures de préemption, soit 39 % des 510 préemptions exercées au total. Cet outil juridique est donc pleinement opérationnel. En outre, qualitativement, la mise en oeuvre de ce droit permet de contrecarrer la tendance au morcellement extrême de la forêt francilienne. Les 198 ventes sur lesquelles la Safer est intervenue représentent une surface totale d'environ 105 hectares de foncier forestier. Il en ressort

L'efficacité du dispositif comporte donc un volet préventif et dissuasif particulièrement utile, et c'est une excellente chose puisque, lorsqu'une parcelle est vendue, illégalement défrichée et artificialisée, il est excessivement difficile pour les communes et les maires d'intervenir, car notre droit prévoit un certain nombre de souplesses permettant de s'installer à titre provisoire dans certains habitats démontables ou mobiles. S'agissant de la conformité juridique de ce texte, qui ne s'applique que sur une portion du territoire hexagonal, on peut citer des précédents, comme la décision du Conseil constitutionnel qui a validé la création d'une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux en Île-de-France. Pour justifier la nécessité d'un dispositif spécifique à la forêt francilienne, il convient de rappeler que celle-ci est trois fois plus morcelée que dans l'ensemble de l'Hexagone, avec des parcelles d'une superficie moyenne d'un hectare, ce qui affaiblit son potentiel de gestion et de protection. Les forêts franciliennes doivent donc rester en mesure de bénéficier de ce que les scientifiques appellent l'effet fertilisant du CO2, qui permet aux arbres de se développer en capturant du carbone tout en diffusant de l'oxygène dans l'atmosphère francilienne. De plus, ces peuplements forestiers sont les garants d'une certaine fraîcheur climatique pour les Franciliens, puisqu'un arbre d'assez grande taille puise environ 100 litres d'eau par jour dans le sol et en vaporise une grande proportion dans l'air. Je précise également ici que, comme l'ont souligné fort justement en commission nos collègues Daniel Gremillet Jackie Pierre, Franciliens d'adoption, il s'agit non pas de mettre la forêt « sous cloche », mais de pouvoir l'exploiter comme elle doit l'être. Le 8 janvier dernier, la commission des affaires économiques, sous la présidence de notre collègue Sophie Primas, a examiné le rapport et adopté sans modification, selon la procédure de législation en commission, cette proposition de loi. L'unanimité étant rare de nos jours, c'est donc avec plaisir et sans réserve que le groupe Les Républicains votera ce texte. Personne ne demande plus

Ce Lorrain éminent avait vu juste en déclarant que l'Europe ne se ferait « pas d'un coup ni dans une construction d'ensemble », mais qu'elle prendrait la voie de « réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait Force est de constater que ce souffle, aujourd'hui, manque à notre continent. L'Union européenne est en panne de projets fédérateurs, sa législation est vécue davantage comme une contrainte que comme une opportunité de développement économique et nos concitoyens peinent à se retrouver dans cet ensemble désormais très vaste. L'Union européenne a d'abord été une réalisation économique, avant de devenir, avec le traité de Maastricht, un ensemble politique sur la voie de l'unification. Notre Union a, par sa taille, par sa force économique et commerciale, par la détermination d'une partie croissante de sa population aussi, tout intérêt à devenir, demain, une puissance écologique de premier plan. Comment le pourrait-elle ? J'identifie, pour ma part, trois axes de travail. Le premier de ces chantiers est d'ordre philosophique. Il s'agit de réconcilier l'écologie et la croissance économique. Certains, depuis longtemps, ont souhaité faire de l'écologie sans la croissance et, parfois, contre Cela a donné les discours les plus rétrogrades, déclinistes et collapsologues. L'avenir de notre planète mérite pourtant d'être abordé avec sérieux et hauteur de vue, grâce à une action éclairée par la vérité scientifique. Héritiers des Lumières, nous devons porter une adaptation de nos sociétés aux nouveaux défis grâce à la raison et au progrès, et non sombrer dans un déclinisme moribond, aux relents populistes. Une écologie privée de croissance, soyons-en sûrs, ne bénéficierait qu'aux éternels donneurs de leçons pour qui la cause environnementale s'est toujours résumée en un « yakafokon » démagogique. Elle ne pourra en revanche que pénaliser ceux pour qui l'écologie a toujours été ressentie comme une contrainte, alors qu'elle aurait dû être source de chances nouvelles. Pour autant, mes chers collègues, soyons lucides : une croissance sans écologie aurait des effets tout aussi néfastes. Les années de prospérité économique reposant sur une production carbonée et polluante sont à oublier, au risque pour les acteurs économiques qui décideraient de maintenir ce modèle de croissance d'être confrontés très prochainement à des pénuries évidentes de matières premières. Le pragmatisme nous commande donc fil des modèles économiques permettant un développement soutenable dans le temps long. les années de « croissance sale » sont à oublier parce qu'une partie toujours plus nombreuse de nos nations n'en veut plus. La revendication climatique a parfois ses excès, et toujours il faudra, dans ces débats complexes, l'appui de la science et de la raison. Pour autant, refuser de constater que les conditions de la croissance ont changé, c'est se condamner à la « cornerisation » politique autant qu'au suicide économique. Ouvrons les yeux : quand quand la France aligne péniblement 100 millions d'euros pour son plan hydrogène, la Chine a déjà investi 11 milliards d'euros ! Bien plus qu'un créneau idéologique, je considère depuis longtemps l'écologie comme une occasion majeure de développement économique, de cohésion sociale et d'interaction territoriale. Le deuxième défi à relever est donc celui de l'unité de notre continent, autour d'une ambition climatique forte. Vous le savez, la France a consenti des efforts importants au nom de la transition écologique. Ces efforts ne seront acceptés que s'ils sont justes et équitablement partagés par tous. Mais si nous sommes les seuls à faire des efforts, nous perdrons le double combat de l'efficacité environnementale et de l'équité économique. Les exemples sont nombreux, dans nos départements, d'entreprises pénalisées par cette absence de réciprocité normative entre États membres de notre Union européenne. Des entrepreneurs se battent pourtant pour accélérer la transition écologique de leurs productions. Comment, dès lors, accepter que, à quelques centaines de kilomètres de là, un membre éminent de l'Union puisse remettre en service ses centrales à charbon ? Comment expliquer qu'un autre État puisse délibérément refuser de s'engager avec le reste de l'Europe sur la voie d'un continent en voie de verdissement ? Comment continuer à imposer une fiscalité carbone aussi élevée dans notre pays, alors que seuls cinq États membres s'en sont dotés ? Je crois, mes chers collègues, que nous ne pouvons plus faire comme si notre pays évoluait en dehors d'une économie ouverte, au sein de laquelle les actions de l'État ont souvent le même effet qu'un éléphant au milieu d'un magasin de porcelaine. L'Union européenne a donc tout à gagner à l'harmonisation des législations environnementales. la France peut être, avec les pays de l'Europe du Nord, une force de transformation. Ne nous y trompons pas : sans revitalisation des secteurs primaire et secondaire, nous ne parviendrons que difficilement à maintenir notre rang dans la mondialisation. Or l'écologie, à condition d'être une ambition partagée par toutes les nations européennes, peut être demain, je le crois, une composante majeure des politiques économiques européennes. Si tous les États membres de l'Union avancent dans la même direction, nous pourrons alors sortir de la dépendance aux importations qui affaiblissent aujourd'hui l'économie de notre continent. C'est notamment vrai pour l'énergie. Qu'attendons-nous pour bâtir une union de l'énergie où tous les pays mettraient en commun leurs avantages comparatifs, après analyse en cycle de vie- de vie- le nucléaire français, le renouvelable pour l'Allemagne ou la biomasse pour l'Europe du Nord -, pour aboutir à une vraie indépendance énergétique Qu'attendons-nous pour donner à la politique commerciale européenne son pendant industriel, avec des investissements massifs dans la transition énergétique, pour une véritable valeur ajoutée à l'international et l'exportation de nouveaux brevets ? Qu'attendons-nous, enfin, pour aligner les standards qualitatifs de l'agriculture européenne sur un mieux-disant environnemental, garantissant tout autant la sécurité sanitaire, la traçabilité et la qualité des produits, pour mettre fin aux importations, qui sont aberrantes sur le plan écologique et destructrices sur le plan économique ? Vous le voyez, mes chers collègues, ce n'est donc que dans la conjugaison des forces et dans le juste partage des efforts, que notre Union européenne pourra apparaître, à la face du monde, comme une puissance économique et écologique unie et cohérente, capable de valoriser le travail de ses entreprises et de ses agriculteurs. C'est aussi la condition pour que nos citoyens retrouvent foi dans le projet européen. En effet, si l'Europe tarde encore à agir pour le climat, elle aura beau être un géant économique, elle n'en restera pas moins un nain Pour que ce chantier que je nous propose ait du sens, il lui faut une clé de voûte, qui constitue le coeur de la proposition de résolution que nous débattons et qui représente la troisième piste de réflexion. Pourquoi une barrière écologique aux frontières de l'Union européenne ? L'enjeu est double. Comme je l'ai indiqué, nous ne pouvons plus accepter que l'écologie soit vue comme une entrave au développement économique de nos entreprises. Or elle l'est encore largement aujourd'hui, à cause de la concurrence déloyale que nous fait subir un certain nombre de nos partenaires commerciaux, affranchis de toutes les règles environnementales que nous avons choisi d'adopter.

Le bilan carbone des économies européennes est aujourd'hui dominé, non par les émissions de CO2 nationales, mais par l'ensemble des émissions liées aux importations. Nous pourrons donc continuellement durcir nos normes, alourdir nos fiscalités énergétiques, si rien n'est fait pour faire changer nos partenaires commerciaux, nous aurons perdu d'avance la bataille du climat. Il convient ainsi de rétablir une justice économique et écologique dans nos échanges, par l'instauration d'une taxation des importations provenant de pays s'affranchissant de tout engagement climatique. C'est tout le sens de la proposition de résolution que nous présentons devant vous,

pour réaliser dès maintenant, alors même qu'un consensus sociétal existe, les évolutions nécessaires à l'échelon de l'Union européenne ; c'est en effet celui qui convient le mieux pour que les actions nationales ne se retrouvent pas prisonnières de l'attitude du passager clandestin adoptée par d'autres pays. L'un de nos illustres prédécesseurs au Sénat, Victor Hugo, avait l'audace de déclarer : « Ce que Paris conseille, l'Europe le médite ; ce que Paris commence, l'Europe le continue. ». Entendez donc, madame la secrétaire d'État, la voix du Sénat, qui vous invite et vous presse d'agir pour réconcilier économie et écologie au service de la prospérité de l'Union européenne et de son rayonnement mondial. Bravo ! La parole

n'a plus droit au chapitre, et c'est une bonne chose. Il faut dire que les événements climatiques extrêmes en France comme dans le monde permettent difficilement d'ignorer l'urgence environnementale à laquelle nous faisons face.

C'est pourquoi il nous semble nécessaire que le sujet de la « barrière écologique aux frontières » soit à l'ordre du jour. J'espère que cette idée, qui figure aujourd'hui dans tous les discours, pourra déboucher sur la mise en place de mécanismes à la fois efficaces et justes. Ce sujet semble, dans son principe en tout cas, faire consensus dans notre pays : la taxation carbone aux frontières faisait partie du programme de la plupart des formations politiques françaises lors des élections européennes. De même, le G, la présidente de la Commission européenne a annoncé envisager un ajustement carbone aux frontières si les écarts entre l'Union européenne et le reste du monde persistaient. En effet, en plus de rétablir une certaine équité dans les échanges internationaux, une taxation bien pensée pourrait inciter les entreprises à adopter des technologies bas-carbone et à apporter les recettes nécessaires au financement

Or on sait qu'il est nécessaire, pour des questions d'acceptabilité, mais aussi et surtout de justice sociale, que la transition écologique contribue à réduire les inégalités.

de résolution prévoit ainsi de taxer aux frontières les produits fortement émetteurs de gaz à effets de serre. Pour être légitime, il faudrait que cette taxe s'applique de manière identique

frontières ne doit pas constituer un simple outil de protectionnisme : il doit favoriser les produits les plus respectueux de l'environnement et inciter l'ensemble des acteurs à faire évoluer leurs pratiques, et pas uniquement les producteurs des pays tiers. L'autre mesure proposée au travers de ce texte, à savoir une taxation des produits provenant de pays ne respectant pas les standards européens en matière environnementale,

Quelle pourrait être la légitimité de la France à exiger un renforcement de la taxe carbone en Europe, alors qu'elle fait partie des plus mauvais élèves européens en matière de recettes fiscales environnementales en pourcentage du produit total d'impôts et de cotisations ? ! Même l'Europe est loin d'être exemplaire concernant sa politique de réduction de gaz à effet de serre. Comme le relevait le Réseau Action Climat à ce sujet, les émissions de l'industrie n'étant pas en baisse en Europe faute de réelles mesures, la proposition d'une taxe carbone aux frontières revient à faire payer notre inaction par le monde extérieur. Pour mener à bien cette nécessaire transition écologique, nous devons de mener une action volontariste, à l'échelon tant national qu'intraeuropéen, pour amorcer un véritable changement de nos modes de productions et de consommation. Pour nous, la nécessaire relocalisation de l'économie ne doit pas seulement passer par une taxe carbone. Ainsi, réserver les marchés publics à des entreprises européennes serait une autre piste pour amorcer une transition. De même, en agriculture, pour citer un secteur particulièrement touché par la compétition mondiale, afin d'éviter que nos paysans ne subissent la concurrence déloyale des pays n'ayant pas les mêmes normes que les nôtres, la relocalisation de l'alimentation- nous aurons l'occasion de revenir très souvent sur ce sujet cette année -, notamment dans la restauration collective, nous paraît une priorité. Par ailleurs, les questions de la responsabilité différenciée des pays du monde dans le réchauffement climatique et de l'impact potentiel de cette taxe sur les pays émergents ne sont pas non plus abordées dans cette proposition de résolution. Or elles doivent être posées. Enfin, les normes environnementales sont présentées ici essentiellement sous l'angle d'une perte de compétitivité. Ce texte n'appelle pas réellement à plus d'ambition nationale.

favorables au commerce international, à condition bien sûr que celui-ci soit régulé. Or les tensions commerciales, pour ne pas dire les prémices de guerre commerciale, que l'on a pu voir émerger ces derniers mois, mais surtout

il agit dans ce sens. On l'a vu avec le CETA, la mise en place de la commission Schubert et la volonté d'assurer un suivi et d'améliorer la prise en compte des enjeux sanitaires et environnementaux ; on l'a vu également lors du rejet du projet d'accord commercial avec le Mercosur,

comme l'un des éléments essentiels dans les accords passés. C'est dans le cas des négociations actuelles entre l'Union européenne et l'Indonésie, mais aussi, plus récemment, cet été, dans les discussions du G7 de Biarritz sur l'Amazonie.

par le Gouvernement, d'un mécanisme d'inclusion carbone aux frontières permet de contourner cet obstacle et le risque d'accusation de protectionnisme.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, avec la nouvelle année, il semblerait que le groupe Les Républicains entame sa transition écologique. En effet, les auteurs du texte qui est soumis aujourd'hui au Sénat ne proposent rien de moins que la mise en oeuvre d'une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, afin, je cite l'exposé des motifs, « d'inciter nos partenaires extraeuropéens à une plus grande exigence environnementale

Par ailleurs, comment comprendre cette initiative, alors même, chers collègues du groupe Les Républicains, que votre groupe parlementaire au Parlement européen, le PPE, a voté tous les traités de libre-échange qui justement suppriment toutes les barrières aux frontières, qu'elles soient financières ou normatives, engageant une régression environnementale et sanitaire très dangereuse, faisant primer les marchés sur les droits humains. Comment comprendre cette prise de conscience ? Il faut sans doute mieux lire la proposition de résolution pour bien saisir votre propos et comprendre que cette proposition d'action résolue à l'échelon européen se conjugue avec l'idée d'un retour en arrière dans les politiques nationales. En effet, vous jugez la taxe carbone nationale injuste et inefficace par nature, dans la mesure où elle pèse sur les entreprises. Voilà votre véritable sujet : il s'agit bien, par cette résolution, d'écarter toute norme et toute fiscalité pour les entreprises nationales.

groupe Les Républicains, compétitivité se conjugue ainsi toujours avec déréglementation, bien loin des préoccupations écologiques, sociales ou démocratiques. L'intérêt de cette proposition de résolution réside donc non pas dans ce qu'elle contient, mais plutôt dans ce qu'elle ne dit pas le refus de toute fiscalité pour les entreprises et de normes environnementales considérées, à tort, comme des handicaps à la compétitivité. On a d'ailleurs rarement vu une proposition de résolution présenter aussi peu de liens avec son objet et sa conclusion. Loin de vous intéresser à l'ambition écologique du continent, vous ne cherchez au fond qu'à retarder les efforts de la France. C'est sans doute d'ailleurs pour cela que vous n'avez pas déposé de proposition de résolution européenne. Mes chers collègues, tout cela reste très « vieille époque » ! Ah ! Nous considérons bien au contraire que les entreprises doivent participer au changement de modèle environnemental. C'est même la manière de les rendre innovantes. Par ailleurs, une taxe carbone nationale n'est pas antinomique avec un quelconque dispositif européen.

Une limite importante tient également au fait que cette fiscalité n'est que très peu fléchée au profit de la transition écologique : elle vient en soutien aux politiques d'austérité, justifiant au passage la régression de la fiscalité sur le travail et sur le capital. C'est d'ailleurs ce qui a soulevé la colère des « gilets jaunes au travers de la proposition de résolution, nous pensons que l'existence de normes environnementales est justifiée et témoigne de la prise en compte d'un intérêt général devenu incontournable : la protection de la biodiversité et du vivant et la préservation des ressources, qui ne sont pas un puits sans fin. Nous notons d'ailleurs que le groupe Les Républicains vote toujours toutes les mesures allant dans le sens d'une régression des normes environnementales, alors même que la situation actuelle nécessite de limiter très fortement les transports, de relocaliser et de diminuer les impacts sur la planète. La dernière phrase de l'exposé des motifs en dit long : « La proposition de résolution, qu'il vous est demandé de voter, porte la volonté d'une vision ambitieuse de l'écologie, facteur de croissance et de développement, au service des intérêts environnementaux et économiques de l'Union européenne. » Le mythe de la croissance infini est tenace et témoigne de l'absence de compréhension des enjeux environnementaux d'une consommation économe des ressources et de sobriété Pour en revenir au fond de votre proposition, nous considérons pour notre part que, si l'idée d'une taxe carbone aux frontières est intéressante, elle est largement insuffisante pour rompre avec un modèle européen libéral. Comment d'un côté instaurer une barrière écologique et de l'autre accélérer tous les politiques de libéralisation des services publics, sont justement de formidables outils de lutte contre la pollution ? Comment affirmer agir pour le développement du fret ferroviaire tout en libéralisant le rail ? Comment promouvoir la production d'une énergie propre en privatisant les moyens de production ? C'est un contresens que de promouvoir d'un côté la protection de l'environnement et, de l'autre, de mener des politiques uniquement tournées vers le profit et la course aux dividendes, des politiques qui accélèrent le pillage des ressources et qui détruisent nos communs Il faut donc, pour accompagner un dispositif bienvenu de barrage écologique aux frontières, dénoncer tous les accords de libre-échange, instaurer à l'échelon européen un haut niveau de garantie pour les services publics et organiser une harmonisation fiscale et sociale pour lutter contre les dumpings environnementaux et sociaux qui s'opèrent au sein même de l'Union européenne.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le mécanisme de barrière écologique aux frontières, dont il est question aujourd'hui, est soutenu depuis le début des années 2010 par la France et les gouvernements successifs. Il vient apporter des réponses concrètes à la réduction nécessaire et souhaitée des émissions de gaz à effet de serre Je tiens à remercier le groupe Les Républicains et les sénateurs Jean-François Husson et Bruno Retailleau, qui nous offrent l'occasion d'approfondir ce sujet devenu fondamental. Ah ! Nous l'avons remarqué lors des élections européennes du mois de mai dernier, l'idée d'une taxe écologique aux frontières de l'Europe a été très largement partagée par le spectre politique en France. de la proposition de résolution le précisent, l'échelon européen semble le plus indiqué pour une efficacité réelle du mécanisme et une protection de nos engagements et de nos règles intérieures. Le gouvernement actuel fait de ce mécanisme d'ajustement aux frontières un point essentiel de sa vision environnementale et économique européenne, ce que nous saluons, tout comme est essentielle l'importance de la réciprocité dans les accords commerciaux que l'Union européenne est amenée à conclure avec le reste du monde. Il s'agit d'un instrument parmi d'autres du respect de notre modèle, de nos règles et de nos valeurs. L'Union européenne a consenti des efforts notables sur ce sujet, grâce à la nouvelle génération d'accords internationaux qui inclut un volet social et environnemental. Nous devons poursuivre notre engagement dans ce sens. Le refus de négocier des accords avec des alliés ne respectant pas nos principes doit être considéré comme une juste affirmation de notre identité collective et une volonté de préserver notre système. L'Europe, qui aspire à la neutralité carbone à l'horizon 2050, est consciente de l'importance d'un mécanisme d'ajustement du carbone aux frontières. La nouvelle Commission européenne l'inscrit d'ailleurs dans la première partie de sa communication présentant son Pacte vert européen. Une proposition sera formulée sur le sujet au cours du dernier trimestre de l'année 2021 ; nous y serons très attentifs et souhaitons que le gouvernement français reste mobilisé sur cet enjeu. La semaine dernière, le commissaire européen Thierry Breton, présentant les grandes lignes de son projet, a expliqué que le travail s'orientait « pour faire en sorte que nos concurrents paient le juste prix des normes en vigueur chez nous ». C'est important pour l'environnement comme pour notre compétitivité. de résolution rappelle que les entreprises vertueuses européennes pourraient être pénalisées par rapport au reste des puissances mondiales. Ces phénomènes de concurrence déloyale et de distorsion ne sont pas acceptables. de carbone, comme on les appelle, profitent de l'absence du mécanisme juste, clair et efficace que nous appelons de nos voeux. De nombreuses questions se posent quant à la forme que pourrait prendre un tel mécanisme. de résolution évoque la taxation de produits importés fortement émetteurs ou de produits provenant de pays qui ne respectent pas les standards européens en matière environnementale. Ce sont des pistes intéressantes, qui pourraient garantir l'efficacité du dispositif. Cependant, des limites et des obstacles devront être surmontés. Tout d'abord, l'Europe doit s'accorder. La vision française de la taxe carbone aux frontières semble s'imposer peu à peu, mais nous devrons trouver des points de compromis. Nous avons noté récemment la complexité des échanges sur la neutralité carbone de l'Union européenne en 2050 et l'absence de participation de la Pologne à ce dispositif, Les questions fiscales relèvent de la compétence nationale, et il faudra obtenir l'unanimité des États membres pour créer une taxe écologique à l'échelon européen. Certains de nos partenaires restent à convaincre. Par ailleurs, comme le souligne très justement la proposition de résolution, la barrière écologique aux frontières devra respecter les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Nous connaissons tous le principe de non-discrimination des produits similaires, d'où la nécessité d'établir le bon format, afin de s'assurer d'une dérogation efficace. Enfin, la dernière interrogation que je souhaite porter à votre attention, mes chers collègues, porte sur la méthode de mesure de l'empreinte des produits et sur le montant du prix du carbone qui seront suffisamment efficaces pour permettre de créer une barrière performante et influente.

Cette taxe pourrait ainsi créer parallèlement deux cercles vertueux : un premier, international, où entreraient le plus de pays possible, qui réduirait notre impact global sur l'environnement ; un second, européen, où la taxe permettrait de financer la transition écologique de notre ensemble.

les moyens financiers se révéleront déterminants. C'est pourquoi il est primordial de redistribuer de manière pratique et utile les recettes d'un tel mécanisme. Le gouvernement français doit continuer à défendre la taxe carbone et à persuader ses partenaires européens de construire un mécanisme performant. Le groupe Les Indépendants en est convaincu et votera donc cette proposition de résolution. Il y va de la protection de notre modèle et de notre compétitivité, mais aussi de l'influence mondiale que l'Europe ambitionne d'avoir sur les sujets économiques et environnementaux dans les décennies à venir. Mes chers collègues, l'horizon 2050 commence aujourd'hui.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, voilà sept mois, la mission d'information sur l'avenir de la sidérurgie présentait son rapport final. Sa conclusion était claire : il est urgent de « donner des armes » aux producteurs français d'acier, face à une compétition mondiale féroce, à des concurrents proposant des prix toujours plus cassés et au défi immense de la transition environnementale. La proposition de résolution qui nous est présentée aujourd'hui répond à l'appel lancé par ce rapport d'information. Elle vise justement à « donner une arme » concrète aux entreprises européennes, afin que l'ambition écologique, qui ne doit pas être remise en question, dépasse les frontières de notre marché intérieur. Dans le cas de l'acier, ressource d'importance stratégique que nous avons étudiée de près, le déséquilibre est flagrant. L'industrie française consomme en majorité de l'acier importé, alors même que nous avons fermé 144 des 152 hauts-fourneaux français en cinquante À l'inverse, la Chine produit aujourd'hui la moitié de l'acier mondial, en grande partie dans des fourneaux obsolètes et extrêmement polluants, mais elle ne connaît ni quota carbone ni taxation énergétique. Le résultat est clair : l'acier plat chinois est en moyenne environ 20 % moins cher que l'acier européen, à qualité et techniques égales. Les importations d'acier par la France ont augmenté de 70 % en cinq ans. Entendons-nous bien : nous risquons là de manquer notre objectif ! Au-delà de notre industrie, c'est la protection de l'environnement qui pâtit de ces déséquilibres. L'empreinte carbone de la France s'est détériorée malgré tous les efforts des acteurs économiques, malgré les immenses efforts financiers consentis. Je rappelle, par exemple, que la « compensation carbone » coûte, à elle seule, 280 millions d'euros par an à notre pays. La transition énergétique et écologique de l'industrie européenne ne pourra se faire si les politiques publiques tuent les entreprises les plus vertueuses. Je partage donc entièrement l'objectif de la proposition de résolution de Jean-François Husson et Bruno Retailleau : il faut restaurer des conditions de concurrence équitables, en compensant le déficit de compétitivité résultant des contraintes environnementales imposées à nos entreprises. Même si ces dernières entreprises doivent disposer des outils adaptés. La bonne solution, c'est d'inciter nos partenaires commerciaux à adopter des modes de production plus vertueux, sous peine d'acquitter une taxe aux frontières de l'Europe.

de défendre auprès des institutions européennes la mise en place d'un mécanisme d'inclusion carbone aux frontières du marché intérieur. Aujourd'hui, la réflexion mûrit, et la dynamique est bonne : la nouvelle Commission a repris cette proposition, émise de longue date par la France. Nous demandons à l'exécutif de poursuivre ses efforts, afin de rallier tous les États membres. Il faut enfin entrer dans une dynamique vertueuse, constructive, concrète, grâce à laquelle les efforts des industriels en faveur de l'environnement seront réellement valorisés, plutôt que d'être vus comme des poids pour l'emploi et la prospérité de l'Europe. En conclusion, madame la secrétaire

remercier notre collègue Jean-François Husson de nous permettre de débattre de la stratégie de l'Union européenne en matière de lutte contre les dérèglements climatiques, de ses conséquences économiques éventuelles et des mesures à adopter pour concilier développement durable, développement économique et inclusion sociale. Aujourd'hui, au travers de cette proposition de résolution, Jean-François Husson lance un appel à la vigilance et à l'action : il s'agit de mettre en oeuvre des mécanismes d'accompagnement adaptés à l'échelon européen. C'est une nécessité, alors que le Conseil européen, suivant le Pacte vert pour l'Europe présenté par la Commission, ambitionne de faire de l'Europe un continent climatiquement neutre d'ici à 2050. L'Europe, qui souhaite être à la pointe de l'action contre les dérèglements climatiques, sera ainsi exemplaire dans la mise en oeuvre de l'accord de Paris faut toutefois pas se voiler la face : atteindre la neutralité carbone demandera d'intenses efforts. La Commission européenne le souligne d'ailleurs dans sa communication sur le Pacte vert, en affirmant qu'il faut « transformer l'économie de l'Union ». Pour mener à bien cette transformation, la Commission entend utiliser de nombreux leviers, que ceux-ci soient budgétaires, fiscaux ou même taxonomiques, pour encourager les investissements

Certaines filières bénéficieront de cette transformation économique. Le développement des technologies bas carbone représente un potentiel considérable. Il y a là une occasion que l'Europe doit saisir en développant des filières à la fois innovantes, compétitives et pourvoyeuses

D'autres filières subiront des contraintes nouvelles, et il faudra les accompagner. Tel sera notamment l'objet du nouveau fonds de transition promis par la Commission. Je forme le voeu que cet accompagnement soit bien calibré, afin d'éviter que certains de nos concitoyens ne se sentent exclus de la marche de l'Europe. L'Europe n'évolue pas dans une bulle, à l'abri des contraintes extérieures. L'émergence sur notre sol de processus industriels vertueux, qui nécessitera des investissements gigantesques, n'aura qu'une portée limitée pour lutter contre le changement climatique si les conditions de l'échange international n'évoluent pas et si nous ne sommes pas en mesure de lutter contre le dumping écologique. Rappelons à cet égard que les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Brésil ou encore la Russie n'ont pris aucun engagement similaire à ceux de l'Europe, et que rien n'indique qu'ils le feront dans un proche avenir. J'ajoute, sans vouloir être provocateur, que

son expertise et ses ressources financières pour inciter les pays de son voisinage et ses partenaires à la rejoindre sur une trajectoire durable », mais aussi qu'elle souligne « la nécessité de préserver sa sécurité d'approvisionnement et de maintenir sa compétitivité, même lorsque les autres ne sont pas disposés à agir ». Ne soyons pas naïfs,

De manière très concrète, lors de sa venue à Paris la semaine dernière, au cours de laquelle il s'est entretenu avec le président Larcher, le commissaire européen au commerce Phil Hogan a indiqué qu'il entendait faire du respect de l'accord de Paris une clause essentielle des futurs accords commerciaux. C'est un point important, qui témoigne de la volonté de cette commission d'affirmer la puissance commerciale de l'Europe et d'utiliser les relations commerciales pour « faire la norme » à l'échelon mondial. Je le dis souvent : la norme fait le marché.

le risque de fuite de carbone, c'est-à-dire la possibilité que des productions soient transférées de l'Union vers des pays moins ambitieux. J'aurais encore beaucoup à dire, mais je serais alors rappelé

Si un mécanisme de compensation carbone devait être instauré, un peu comme celui qu'envisage la Commission européenne, comment traiterions-nous alors les grandes industries qui, aujourd'hui, bénéficient de quotas gratuits jusqu'en 2030 ? Devraient-elles aussi payer ?

de continuer à commercer, comme si de rien n'était, avec des pays qui ne respectent pas l'accord de Paris. Nous devons utiliser la force et la taille du marché européen pour inciter nos partenaires à le respecter. Il faut

? De ce point de vue, la Chine, qui a mis en place, je le rappelle, un marché carbone, peut être un partenaire de travail sur ce type de certification. Il faut savoir que si l'on vise les grandes industries émettrices de carbone,

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier le groupe Les Républicains de cette proposition de résolution, qui est cohérente avec l'actualité européenne récente et qui défend une certaine vision européenne, sur laquelle je reviendrai. En effet, la nouvelle Commission européenne souhaite renouer avec un agenda positif, avec un agenda positif, l'objectif étant de faire de l'Union européenne le premier continent neutre en carbone en 2050, grâce à la mise en oeuvre de plusieurs politiques d'envergure, telles qu'un plan d'investissement massif dans la transition écologique ou encore la création d'une taxe carbone aux frontières. Ce projet pourrait être vu comme le nouvel acte protectionniste d'une guerre commerciale, qui reléguerait la lutte contre le changement climatique derrière des intérêts nationaux. Il n'en est rien Au contraire, un tel outil permettrait enfin à l'Union européenne de se doter d'une stratégie d'ensemble et de concilier ambition écologique et efficacité économique. Jusqu'alors, les gros émetteurs participaient à un marché européen des quotas de carbone, qui a rapidement perdu sa crédibilité et qui a envoyé des signaux économiques contradictoires. Les émetteurs diffus, quant à eux, étaient soumis à des taxes nationales sur le carbone, taxes non coordonnées, voire concurrentes. Or une taxe aux frontières permettrait, d'une part, de prévenir les fuites de carbone, qui rendent les dispositifs nationaux inefficaces, et, d'autre part, de protéger les entreprises européennes contre tout risque de concurrence déloyale de la part d'acteurs non soumis aux mêmes contraintes. Si l'Europe veut être pionnière dans la transition écologique, elle devra poursuivre une politique climatique ambitieuse consistant à restaurer la crédibilité du marché du carbone en interne, et mettre en place la taxe carbone aux frontières, afin de compenser l'impact du prix du carbone sur la compétitivité des entreprises européennes. La transition La transition écologique ne doit pas opposer écologie et compétitivité ; elle ne doit pas non plus opposer écologie et justice sociale. À cet égard, l'objectif des taxes nationales reste bien de verdir la fiscalité, et non de l'alourdir. De même, une fiscalité carbone aux frontières aurait des effets redistributifs plus importants qu'une taxe carbone domestique, en ce qu'elle porte sur des biens substituables, contrairement aux produits énergétiques. En parallèle, les objectifs du imposent de soutenir les investissements dits « verts ». À cet égard, je suis convaincu de la nécessité de faciliter de tels investissements, en permettant aux États membres de les extraire du pacte de stabilité et de croissance, comme l'a suggéré récemment le nouveau commissaire à l'économie, Paolo Gentiloni. C'est une position que je partage pleinement, pour l'avoir suggérée dans une proposition de résolution déposée au Sénat le 10 septembre dernier. Je le disais en introduction, la taxation du carbone aux frontières de l'Europe n'est pas une manière pour l'Europe de défier ses partenaires commerciaux. Alors qu'un prix du carbone n'a pas pu être inscrit dans l'accord de Paris, la mise en place de cette taxation au sein de l'Union européenne assurerait au continent une crédibilité sur la scène internationale et une influence sur ses partenaires. Elle traduirait également un pouvoir d'initiative retrouvé, qui permettra à l'Europe, j'en suis sûr, d'orienter les grandes transformations que connaît notre monde et de montrer, à rebours du constat amer de Paul Valéry, qu'elle est capable d'avoir « la politique de sa pensée ». La parole

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la contradiction est éternelle entre la croissance économique, la nécessité d'être compétitifs et l'urgence écologique. À l'heure de la nécessaire mobilisation face aux changements climatiques, tout l'enjeu est de rééquilibrer la mondialisation et de réapprendre à produire ce que nous consommons. Nous devons refuser de vivre dans ce monde absurde où on pêche du poisson en Norvège, où on le traite en Chine et où on le consomme en Europe Avec un marché de 500 millions d'habitants comme l'Europe, je suis convaincu que nous pouvons apporter au monde l'équilibre dont il a besoin. Le mathématicien et philosophe Olivier Rey a publié une excellente tribune la semaine dernière. En voici quelques La vérité, c'est que le mondialisme ne peut être la solution à la crise qu'il engendre. Non seulement cela, mais le " no-borderisme ", c'est-à-dire la non-frontière, constitue l'exact inverse de la voie à suivre. Bien sûr, certains problèmes sont globaux. Mais c'est la perte de la mesure locale qui les a engendrés, et c'est recouvrer cette mesure qui peut seule permettre d'y faire face La barrière écologique aux frontières de l'Union européenne que prévoit cette proposition de résolution peut être l'une des solutions pour recouvrer cette mesure locale, qu'elle soit nationale ou européenne.

Nous croyons à l'échange, à la force de nos entreprises, à la compétence de nos agriculteurs et à l'excellence de leurs savoir-faire, mais pour que cette liberté d'échanger ait un sens, il faut que les règles soient les mêmes pour tous La mise en place d'une barrière écologique à l'entrée du marché unique permettrait de remettre de l'équité et de la réciprocité dans les échanges internationaux.

Aujourd'hui en effet, nous trahissons nos industries et nos agriculteurs en faisant entrer en France ces produits internationaux en Europe. Nous créons nous-mêmes la concurrence déloyale ne pouvons continuer à déstabiliser ceux qui produisent chez nous et à encourager ceux qui produisent à l'extérieur, c'est-à-dire ceux qui ne respectent pas les normes environnementales que nous nous fixons.

Il est impensable que l'Europe finance seule la transition écologique. Dans l'espace européen, la France ne représente que 1,2 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

sur un sujet ô combien stratégique, tant pour notre économie que pour le climat. Toutefois, avant d'aller plus avant, permettez-moi de formuler un point de sémantique, car les termes employés, aussi bien dans l'exposé des motifs que dans la résolution elle-même, tendent à brouiller l'objet de la proposition.

mais pourquoi ne pas parler plus distinctement à nos concitoyens et évoquer plus précisément la mise en place d'une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne ? Car c'est bien de fiscalité écologique qu'il s'agit. Nous avions nous aussi soutenu cette idée lors des élections européennes. Le levier écologique constitue aujourd'hui l'outil fondamental pour modifier profondément le fonctionnement de l'Union européenne et permettre à cette dernière de répondre aux demandes de protection et de compétitivité de nos concitoyens et de nos entreprises. Cette nouvelle politique commerciale doit être un outil au service de la transition écologique et climatique, conformément à nos objectifs de neutralité carbone. L'Union européenne doit se saisir de cet outil, aussi bien pour réguler ses importations que pour contraindre par la norme ses partenaires commerciaux.

En clair, il s'agirait de demander à tout importateur d'un produit soumis au système communautaire d'échange de quotas d'émissions, quand il est produit en Europe, de se plier aux mêmes règles européennes que ses concurrents. Le très sérieux Conseil des prélèvements obligatoires confirme, dans un rapport rendu en septembre dernier, que « les initiatives visant à doter l'Union européenne d'un mécanisme de protection commerciale à l'encontre des territoires non coopératifs

L'étude pose bien la question des émissions importées dans notre empreinte carbone et la difficulté d'établir une comptabilité carbone fiable, fidèle à la réalité du processus de production. Cette part de gaz à effet de serre cachée de notre consommation constitue « un angle mort de la lutte contre le réchauffement climatique », qui, de surcroît, ne permet pas de mettre en valeur les efforts des États européens pour réduire leurs émissions. Ainsi, pour la France, indique la même étude, « la diminution constatée des émissions liées à la production nationale depuis plus de quinze ans s'est accompagnée par une hausse continue de celles provenant des importations. L'empreinte carbone des Français en 2015 serait ainsi équivalente à celle de 1995 [et] les émissions importées sont supérieures à celles issues de la production intérieure destinée à la consommation domestique. Ces conclusions justifient l'instauration d'un système de rééquilibrage fiscal aux frontières et démontrent qu'une redistribution totale et progressive du produit de cette taxe aux ménages permettrait d'éviter certains des écueils ayant conduit à la crise des « gilets jaunes

alors qu'elle me semble être au coeur de l'acceptabilité sociale d'une nouvelle prise en compte de l'empreinte carbone de nos échanges, que sa mise en oeuvre soit nationale ou européenne. C'est une part du destin économique et politique de la construction européenne qui se joue au travers de la mise en place ou non de cette taxe carbone aux frontières. Espérons que cette taxe ne connaîtra pas le même sort que la taxe européenne sur les transactions financières, la fameuse taxe Tobin, ou encore que le « veto climatique », qui devait être intégré dans le CETA. Mercredi dernier, la présidente de la Commission se serait rangée à l'idée d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Celui-ci viserait en priorité les secteurs de l'acier, du ciment, du papier-carton, du verre et de la chimie et permettrait de lutter contre la concurrence déloyale- le dumping écologique -, mais aussi contre la tentation pour les entreprises européennes de transférer leur production, et donc le carbone, hors de l'Union

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, dans la fable de l'élu et du citoyen, la morale reprocherait sans doute au politique de prendre des engagements qu'il ne pourra vraisemblablement pas tenir et à ses administrés de croire naïvement à certaines promesses dont ils subodorent pourtant l'infaisabilité. En matière d'écologie, il faut bien l'admettre, on bat des records depuis quelque temps ! À grand renfort de communication, pour ne pas dire de pression,

Depuis Rio, en 1992, les grands sommets internationaux débouchent avec plus ou moins de succès sur des traités dont l'ambition n'a d'égale que l'absence de sanction envers les pays signataires qui ne respecteraient pas leurs engagements, ou même qui y renonceraient totalement, comme nous l'avons vu récemment avec les États-Unis. Même lorsque certains accords, tels que celui de la COP21 à Paris, sont quasi unanimement salués pour l'adhésion générale qu'ils ont suscitée, les moyens financiers engagés ne sont pas à la hauteur, loin de là, et ne sont en vérité jamais quantifiés de manière sincère. Pourtant, personne ne peut croire que l'on va raser gratis, ni qu'une baguette magique sauvera la planète. Rappelons que la France ne compte que pour 1 % des émissions carbone dans le monde, ce qui correspond presque à sa part de population. Cela signifie, compte tenu de nos modes de vie très très énergivores, que notre production énergétique est très largement décarbonée, essentiellement en raison d'une filière nucléaire spécifique à notre pays, n'en déplaise à certains Aujourd'hui, selon les estimations, un habitant de la planète produit entre 5 et 6 tonnes de CO2 par an. À part ceux qui considèrent leurs oeillères comme un guide efficace de réflexion, chacun prend conscience que ce rythme de progression n'est plus supportable, surtout si l'on prend en compte la démographie galopante et l'aspiration au développement, avec pour conséquence une augmentation des besoins énergétiques, tant en Afrique qu'en Asie.

D'autres restent tout simplement sourds à ces préoccupations, qu'ils considèrent comme très éloignées des leurs. Par exemple, quand le Premier ministre norvégien vient parler énergies renouvelables au président polonais, c'est un peu comme si un élu de Maine-et-Loire évoquait le processus de création des communes nouvelles avec un homologue corse lors, que pouvons-nous faire concrètement pour limiter notre production de CO2 et engager une convergence internationale qui ne se traduirait pas uniquement par de beaux discours ? Comment faire comprendre que, si nous ne faisons rien aujourd'hui, nous prenons le risque de franchir un point de rupture irrémédiable ? Comment ne pas faire porter l'indispensable changement des comportements uniquement sur les ruraux, qui devraient répondre aux injonctions d'ultra-urbains habitués au métro, du moins quand les conducteurs de la RATP ne sont pas en grève Conscients de la faiblesse de la portée de chaque action nationale, nous devons user de la masse critique de l'Europe pour peser efficacement face aux géants mondiaux, au niveau tant de la consommation d'énergie que des émissions carbone.

à la présentation par la Commission européenne de son projet de pacte vert pour l'Europe. Le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité apparaissent désormais comme des enjeux existentiels, et nous avons besoin d'une mobilisation transpartisane pour y faire face.

l'impression générale, la COP25 a été décevante. Nouvelle étape de la mobilisation internationale pour la lutte contre le changement climatique, elle devait être celle de l'action, de l'urgence à agir. Mais elle a été bloquée et, sans consensus, les dernières règles relatives à la mise en oeuvre de l'accord de Paris n'ont pu être adoptées. Je modérerais toutefois ce pessimisme en rappelant que c'est aussi pendant cette COP,

Son système d'ambitions croissantes, qui respecte la souveraineté des États, doit nous amener, dès 2020, lors de la COP26 de Glasgow, à présenter des plans nationaux plus ambitieux.

et ensemble. Comme le disait Valérie Létard, c'est un test de crédibilité, d'efficacité, de souveraineté, donc de réactivité. Nous le voyons en effet chaque été, avec des canicules plus longues et plus fortes dans nos villes : les Français et les Européens souffrent. Nous voyons des feux de forêt toujours plus étendus, comme le montrent les spectacles apocalyptiques venant dernièrement d'Australie, mais aussi d'Amazonie, de Californie ou de Scandinavie. aussi la fonte des pôles et la réduction des glaciers sur nos montagnes, la récurrence accrue des inondations, l'accroissement de la puissance et des zones d'activité des tempêtes et des typhons, dont souffrent nos territoires d'outre-mer, ou encore la montée des eaux, lente, mais inexorable, qui ronge nos côtes.

Le Conseil européen s'est mis d'accord en décembre dernier sur un objectif de neutralité pour 2050. L'Europe serait ainsi le premier continent neutre en carbone.

cet objectif est d'ores et déjà inscrit dans la loi française, et je vous remercie, mesdames, messieurs les sénateurs, du soutien que vous nous avez apporté. C'est un succès qu'il convient désormais de consolider, en accompagnant les régions qui seront les plus touchées économiquement et socialement

est la volonté de la France pour le prochain cadre financier pluriannuel, avec comme ambition que 30 % du prochain budget de l'Union européenne soit dédié au climat, et que 10 % soient dédiés à la protection de la biodiversité et à la lutte contre la pollution.

Nous souhaitons en effet que ce pacte vert européen aboutisse à de nouvelles propositions législatives dans les meilleurs délais, afin que ses objectifs soient rapidement atteints. Nous sommes en particulier satisfaits que la Commission ait repris, comme vous le faites dans ces murs, mesdames, messieurs les sénateurs, l'idée d'un mécanisme d'inclusion carbone aux frontières, et que notre proposition visant à faire de l'accord de Paris une clause essentielle des accords commerciaux ait été retenue.

couché sur le papier. Nous devons désormais poursuivre les efforts vis-à-vis de nos partenaires européens. Ils sont certes nombreux à nous faire part de leur intérêt à travailler à l'élaboration d'un tel outil, mais ils se posent également des questions légitimes. Nous devons les rassurer,

l'aluminium, le ciment, et peut-être aussi le papier ou le verre, autant de biens dont nous connaissons les lieux de production et pour lesquels nous pouvons avoir des informations fiables sur leur contenu carbone.

le marché ETS européen aux importations. Nous restons donc dans un domaine de souveraineté. Nous avons mis en place un marché ETS européen et nous souhaitons désormais que le prix

Si nous investissons autant d'efforts dans la mise en oeuvre d'un tel mécanisme, c'est parce que celui-ci constitue une composante essentielle de la politique climatique ambitieuse portée par la France. C'est un enjeu de souveraineté économique. En effet, pour parvenir à la neutralité climatique en 2050, nos entreprises et nos citoyens, partout en Europe, vont devoir fournir des efforts importants,

il faut que les mêmes efforts soient demandés à tout le monde. Tel est l'objet de ce mécanisme d'inclusion carbone aux frontières : faire en sorte que les importateurs payent autant que les producteurs européens, pour une même quantité d'émissions. Ce mécanisme aura également un effet incitatif

pour une réunion avec mes homologues danois, suédois et finlandais, afin de poursuivre le travail et d'élargir la coalition de ceux qui veulent non seulement travailler sur le sujet, mais également le soutenir et s'assurer de sa mise en oeuvre.

l'Union européenne, les États-Unis et le Japon sur le sujet chinois, sur les subventions industrielles et sur la propriété intellectuelle. Cela montre bien que, sur certains dossiers, la persévérance paye. J'espère que nous aurons également, sur ces enjeux de climat, des résultats dans les années qui viennent. D'ici à la COP26 de Glasgow sur le climat, d'ici à la COP15 de Kunming sur la biodiversité, en nous appuyant sur la détermination européenne et sur notre détermination nationale, nous concentrerons nous concentrerons nos efforts pour convaincre les principaux émetteurs de gaz à effet de serre, qui sont aussi les principales forces économiques réunies au sein du G20, de répondre à cette ambition consistant à fixer un prix du carbone au niveau international. Dans ce contexte, vous l'avez compris,

j'espère pouvoir échanger avec vous plus en détail, au fur et à mesure que les négociations européennes sur ces sujets concrets, tangibles et extrêmement importants pour nos territoires se poursuivront. La discussion

et accessible à tous afin de préserver l'activité des entreprises alimentaires françaises, présentée par M. Daniel Gremillet et plusieurs de ses collègues (proposition n° 138, texte de la commission n° 215, rapport n° 214). Dans la discussion générale, la parole est à M. Daniel Gremillet, auteur de la proposition de loi. Monsieur

Cette démarche innovante revient finalement à l'essence même du rôle du Parlement : adopter des lois et en évaluer les effets pour, au besoin, proposer les correctifs nécessaires. En octobre dernier, le groupe de suivi a produit un rapport d'information dressant un premier bilan de la loi Égalim, un an après l'adoption de cette dernière. Ce travail important, réalisé après des auditions effectuées auprès des administrations, des organismes professionnels, professionnels, mais aussi- ce point est important -des acteurs de terrain, a permis de dégager des premières tendances inquiétantes. Bien sûr, il est trop tôt pour tirer des enseignements définitifs sur les effets de cette loi ; ainsi, le titre I organise une expérimentation de deux ans qui est en cours. Au terme de ce délai, nous y verrons plus clair et nous ne manquerons pas d'en tirer les conséquences. Toutefois, les auditions du groupe de suivi ont déjà mis en lumière trois problèmes majeurs posés dès à présent par la loi.

Si les failles sont d'ores et déjà identifiées, il est de notre responsabilité d'agir. C'est en tout cas la position du groupe de suivi qui a déposé, dans la foulée, une proposition de loi comprenant trois mesures d'urgence. Le texte qui est soumis à notre examen aujourd'hui a été signé, à ce stade, par cent quarante-six sénatrices et sénateurs de la quasi-totalité des groupes politiques. Cette Cette capacité des élus à se rassembler autour de ce texte, quels que soient les clivages, est une démonstration de l'intérêt stratégique des sujets évoqués. Monsieur le ministre, c'est de la politique au sens noble du terme, et je souhaite remercier l'ensemble des sénatrices se sont associés à cette démarche. Le Sénat joue son rôle de contrôle de l'action du Gouvernement et est une force de proposition pour améliorer l'efficacité des politiques publiques- c'est essentiel La première mesure proposée dans le texte concerne l'encadrement des promotions en volume. Nous sommes dans le cas d'une disposition rigide qui ne prend pas en compte les réalités très différentes selon les entreprises, les filières, les secteurs. cela pose des difficultés, notamment pour les fabricants de produits achetés par le consommateur de manière impulsive ou pour les producteurs de denrées saisonnières. Pour les entreprises le soutien promotionnel est essentiel. Quand un consommateur ne programme pas son achat à l'avance- c'est le cas pour des produits comme la viande de lapin ou le saumon fumé -, il revient à l'industriel de le convaincre, dans les linéaires, d'acquérir son produit

L'encadrement des promotions limite le volume des ventes. Les résultats sont clairs : les chiffres d'affaires des entreprises concernées se sont effondrés depuis un an. Ils parlent

Et ce qui est le plus paradoxal, c'est que la loi déstabilise les filières qui rémunéraient le mieux les producteurs, des filières qui avaient instauré une indexation des prix avec l'amont agricole. Monsieur le ministre,

La proposition de loi entend remédier à ce problème, en prévoyant de sortir les produits au caractère saisonnier marqué de l'encadrement des promotions en volume. Surtout, j'insiste sur ce point, la mesure ne remet nullement en cause l'esprit de l'expérimentation. Monsieur le ministre,

Ce n'est pas ce type de disposition de bon sens qui est de nature à relancer la guerre des prix dans les grandes surfaces ni à remettre en cause l'expérimentation en cours. En revanche, elle permettrait de sauver

Tous sont aux abois du seul fait de la loi. Il y a un vrai caractère d'urgence. Si le seul contre-argument est celui de ne pas vouloir fausser statistiquement l'expérimentation, permettez-moi, monsieur le ministre, d'en appeler à votre pragmatisme. Des centaines, voire des milliers d'emplois sont en jeu La proposition de loi comporte une deuxième mesure, qui est expérimentale. Cela fait plusieurs années que nous débattons du manque d'efficacité de la renégociation des contrats entre un fournisseur et son distributeur en cours d'année en cas de choc conjoncturel sur le cours d'une matière première. La clause de renégociation ne fonctionne pas, car, une fois activée, tous les points du contrat peuvent être renégociés, ce qui avantage considérablement le distributeur. le texte d'expérimenter la mise en place, dans les contrats, d'une clause de révision automatique des prix, déterminée par les parties, qui s'activerait en cas de variation importante du cours de la matière première principale et fortement présente dans un produit alimentaire. Ce serait par

la proposition de loi que l'ordonnance sur la réforme du droit coopératif publiée par le Gouvernement ne respecte pas le champ de l'habilitation donnée par les parlementaires. C'était le seul point d'accord constaté en commission mixte paritaire entre les deux chambres : plutôt que de signer un chèque en blanc au Gouvernement, les deux chambres ont restreint strictement le champ de l'habilitation. Constatant sans doute que cette habilitation l'empêchait désormais de faire ce que bon lui semblait, le Gouvernement a eu recours à une autre ordonnance pour passer en force Sans même parler du fond de la mesure qui mériterait un débat sur le modèle coopératif, débat dont le Parlement a été privé lors de l'examen de la loi Égalim, il a semblé aux membres du groupe de suivi que le Parlement devait se montrer intransigeant sur le respect des champs d'habilitation qu'il déterminait lorsqu'il confiait au Gouvernement le droit de prendre une ordonnance. C'est pourquoi la proposition de loi ratifie l'ordonnance sur le modèle coopératif corrigée de la partie qui a excédé le champ de l'habilitation. Cette mesure répond avant tout à une logique institutionnelle de défense des droits du Parlement. Si le Gouvernement tient à cette disposition, qu'il la présente dans un projet de loi pour que le Parlement ait enfin le droit de débattre sereinement de nos coopératives agricoles ! Pour conclure, vous l'aurez compris, cette proposition de loi n'a pas l'ambition de résoudre l'ensemble des défis posés à notre agriculture. Elle n'a pas non plus la prétention de revoir l'intégralité de la loi Égalim. Elle entend simplement en corriger les premières failles, car ces dernières posent déjà de graves difficultés dans nos territoires. C'est notre rôle constitutionnel d'évaluer la loi, et le groupe de suivi a voulu mettre ce rôle en avant. Nous sommes donc loin d'une remise en cause politicienne de la loi Égalim adoptée il y a moins d'un an. Au contraire, malgré nos doutes, il me semble que cette proposition de loi entend préserver toutes ses chances d'améliorer le revenu de nos agriculteurs. Enfin, je tiens à remercier Michel Raison et Anne-Catherine Loisier qui étaient rapporteurs

il ferait tout pour qu'elle permette au mieux d'améliorer le revenu agricole. C'est dans cette perspective que nous avions proposé la création immédiate d'un groupe de suivi des effets de la loi pour pouvoir au mieux accompagner son déploiement. Nous avons toujours fait part de nos inquiétudes sur un texte qui nous semblait déséquilibré et qui était loin d'être la loi agricole attendue dans nos campagnes. Comment aurait-il pu l'être, alors qu'il n'agissait que sur les relations contractuelles entre l'agriculteur et ses acheteurs, ce qui représente moins d'un cinquième des recettes Dans le même temps, la France ne mène pas forcément les combats essentiels sur le budget de la politique agricole commune (PAC) ou sur les exportations alimentaires À la lecture de la loi finalement adoptée, nous avions une certitude : elle représenterait une hausse de charges pour les agriculteurs. En échange, le mécanisme du ruissellement contenu dans le texte était loin d'assurer une revalorisation certaine des revenus des agriculteurs en l'absence d'instrument le garantissant. J'ai indiqué à plusieurs reprises que, pour faire ruisseler de l'aval vers l'amont, il fallait une bonne pompe de relevage Tout reposait sur un mot : la confiance entre les acteurs ou, en d'autres termes, la « morale ». Les premiers résultats des négociations commerciales sur les contrats annuels de 2019 ne nous ont pas démentis : la déflation est toujours présente. Hormis quelques emblématiques contrats laitiers, rien n'a changé ! L'argument selon lequel ces éléments ne sont pas représentatifs, car les textes d'application de la loi n'étaient pas tous en vigueur, est insuffisant. De son côté, la grande distribution a bien récupéré bien récupéré les fruits de la hausse du seuil de revente à perte (SRP), mais plutôt que de les redistribuer par une revalorisation des prix accordée à ses fournisseurs, elle a adapté, comme à chaque fois, son modèle à cette nouvelle donne pour limiter l'augmentation des prix pour le consommateur. La hausse du SRP aura servi, cette année, à déplacer la guerre des prix. Elle n'est pas terminée sur les produits des grandes marques et s'est intensifiée sur les produits sous marques de distributeurs (MDD) et dans les rayons non alimentaires. C'est seulement à titre résiduel que le SRP a permis de revaloriser quelques contrats laitiers emblématiques. Cette réalité risque, hélas, de se reproduire en 2020, en dépit de la publication des textes d'application.

aucune information statistique fiable sur les résultats des négociations relatives aux produits MDD. Dès lors, comment mesurer finement les effets de la loi ? À moyen terme, le groupe de suivi poursuivra ses travaux, mais le rapport d'information que nous avons rendu le 30 octobre dernier a démontré que la loi posait des problèmes à court terme. La présente proposition de loi entend, modestement, en limiter les effets les plus néfastes, en comportant trois mesures d'urgence. Tout d'abord, la loi Égalim ne réduit en rien l'exposition des industriels de l'agroalimentaire à la volatilité des prix des matières premières sur les marchés mondiaux. Ils sont le plus souvent pris en étau entre une hausse des prix des denrées agricoles payés aux agriculteurs qui suivent les cours mondiaux et un prix de vente au distributeur très difficilement renégociable. La clause de renégociation des prix ne fonctionne pas bien et la loi Égalim n'est pas allée assez loin sur ce point. Les difficiles renégociations qui ont eu lieu en 2019 malgré la flambée du cours du porc, par exemple, l'ont démontré. C'est la compétitivité de nos entreprises qui est en jeu.

une telle expérimentation sur quelques produits comme la charcuterie ou les pâtes alimentaires ? C'est le pari que fait l'article 2 de cette proposition de loi. Un autre problème posé par la loi est l'assimilation d'une relation entre un associé coopérateur et sa coopérative à une relation entre un fournisseur et son client. Daniel Gremillet en a parlé, les coopératives ne sont pas régies par les mêmes règles que les entreprises privées. Il faut toujours garder à l'esprit cet élément, car les coopératives appartiennent aux agriculteurs ; elles sont le prolongement de leur exploitation et sont, en cela, des acteurs essentiels du monde agricole. Je rappelle aussi qu'une coopérative est une sorte de service public : comme le facteur qui doit distribuer le courrier partout, la coopérative doit ramasser les produits des exploitants partout.

Cela ne veut pas dire que les coopératives doivent être exonérées de toute obligation et que la loi Égalim ne leur est pas applicable. L'ordonnance fait actuellement l'objet d'un contentieux, le juge administratif rendra son verdict, mais en tant que rapporteur du projet de loi Égalim réaffirmer que, dans l'esprit des parlementaires, le champ de l'habilitation ne comportait pas cette mesure. Le rapporteur de l'Assemblée nationale partage ce point de vue. J'en viens, enfin, à la troisième difficulté qui est liée à la rigidité de l'encadrement des promotions en volume pour les produits saisonniers et festifs. Daniel Gremillet a cité les chiffres inquiétants de l'évolution des ventes de certains produits. Permettez-moi d'évoquer des cas concrets

vouloir accorder des dérogations, mais la sécurité juridique est insuffisante, puisque cette possibilité n'est nullement prévue par l'ordonnance. Le seul moyen de sortir ces entreprises de l'ornière, c'est de modifier l'ordonnance dès aujourd'hui pour ôter de l'encadrement des promotions en volume, et non en valeur,

Son adoption ne résoudra pas tous les problèmes posés par la loi Égalim, mais elle réduira certains effets de bord et sauvera,

Cette décision a été prise par l'ensemble de la profession agricole et des acteurs économiques et politiques. Lors du dernier comité de suivi des négociations commerciales,

vous proposez d'expérimenter l'introduction d'une clause de révision des prix, à la hausse comme à la baisse, pour les produits composés à plus de 50 % d'un produit agricole, tout en prévoyant des amendes administratives en cas de non-respect. Le contenu précis de cette clause sera défini par les parties au contrat. La loi a renforcé la clause de renégociation en raccourcissant le délai d'un mois et en obligeant à avoir recours au médiateur des relations commerciales agricoles en cas d'échec. Votre proposition ouvre de nouveau un débat, que nous avions eu dans cet hémicycle, à l'époque où j'étais sénateur, durant l'examen du projet de loi Égalim en première lecture. lecture. Un amendement visant à introduire le même mécanisme avait alors été adopté, contre l'avis du Gouvernement et de mon prédécesseur. Aujourd'hui, la réponse du Gouvernement est identique. Les acteurs économiques, même ceux qui ont des difficultés, nous demandent une stabilité du cadre juridique. Il me semble préférable d'appliquer les dispositions introduites par la loi Égalim, promulguée en 2018, en matière de clause de renégociation et de ne pas bouger maintenant les curseurs. Je crois savoir que cette clause de renégociation a été activée pour les produits charcutiers en 2019. Bien sûr, je le concède, cette renégociation ne va jamais assez vite,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui la proposition de loi modifiant la loi Égalim. de loi fait suite à l'adoption par la commission des affaires économiques du rapport d'information de MM. Daniel Gremillet, Michel Raison et Mme Anne-Catherine Loisier. Je tiens en cet instant à leur rendre hommage pour le travail pertinent accompli. le rapport d'information est critiqué le manque d'efficacité de la loi Égalim concernant la revalorisation du revenu des agriculteurs et sont dénoncés les effets pervers de deux mesures : le relèvement du seuil de revente à perte et l'encadrement des promotions. La loi Égalim a prévu une expérimentation de deux ans concernant ces deux mesures. Je rappelle que les décrets d'application sont sortis en février dernier, il y a moins d'un an. Mes chers collègues, nous devons prendre le temps nécessaire pour tirer les conclusions de ces mesures. L'agriculture s'inscrit dans le temps long. Et comme le rappelle le rapport d'information, la part des recettes des agriculteurs liée aux ventes en grande distribution ne représente qu'une petite partie du revenu de ces derniers. Nous ne pouvons pas obtenir de résultats spectaculaires en si peu de temps. Toutefois, la loi aura eu le mérite de mettre fin à cinq années consécutives de déflation des prix alimentaires. Il est aujourd'hui difficile de faire le bilan si peu de temps après sa promulgation. Comme nous Comme nous avons pu l'observer dans nos territoires, le rééquilibrage des relations commerciales entre producteurs, industriels et distributeurs n'est bien évidemment, pour l'instant, pas satisfaisant. Le constat est toujours le même : l'agriculteur ne vit pas dignement de ses activités. Les PME apparaissent comme les grandes perdantes de la loi. Nous avons constaté une baisse significative de la croissance des produits de grande consommation et des produits frais en libre-service, affectant en particulier les PME. Celles-ci, qui, hier, tiraient le marché, ont brutalement vu leur activité chuter. Ce coût d'arrêt à la croissance des PME est préoccupant. Seules les marques de distributeurs, dont 80 % des ventes sont réalisées par des PME, TPE et ETI, arrivent à tirer leur épingle du jeu. Bien que ce constat soit alarmant, la croissance des PME est affectée par une multitude de mécanismes. Par exemple, ces entreprises ont aujourd'hui de moins en moins le monopole des produits locaux, bio ou sans gluten, qui tirent la croissance. Nous savons que les grands groupes se positionnent de plus en plus sur ces secteurs de marché. Mes chers collègues, les négociations commerciales en cours sont un véritable test. Nous pourrons faire le bilan seulement à l'issue de l'expérimentation du relèvement du SRP et de l'encadrement des promotions. Aussi, le groupe La République En Marche s'abstiendra.

mes chers collègues, que j'avais qualifié le projet de loi Égalim lors des débats au Sénat. Un an après la promulgation de la loi, le constat est unanime : celle-ci est en deçà des aspirations exprimées lors des États généraux de l'alimentation. Elle n'a pas répondu à son premier objectif : un meilleur partage de la valeur et l'assurance d'un revenu décent aux agriculteurs. Le rééquilibrage des négociations commerciales est un échec. L'interdiction des prix de cession à des montants abusivement bas est inopérante. La hausse du seuil de revente à perte et l'encadrement des promotions dans les grandes surfaces ont eu un effet rebond pénalisant pour les PME du secteur agroalimentaire, qui ont vu un net recul de leur chiffre d'affaires depuis la mise en oeuvre de la loi. Comme les autres années, les négociations commerciales de 2019 se sont déroulées dans un climat tendu et restent extrêmement déséquilibrées : chantage aux prix bas, menace de déréférencement des produits, baisse générale des prix d'achat de la grande distribution aux fournisseurs, non prise en compte du prix de revient calculé par les organisations de producteurs. Telle est la réalité de ces négociations qui n'en ont que le nom ! Jamais les promesses de la grande distribution, sur lesquelles les grandes orientations de la première partie du projet de loi étaient fondées, n'auront autant été bafouées. Pendant ce temps-là, le désarroi agricole est toujours aussi profond ; les agriculteurs continuent de vendre à perte leurs productions quand les marges de l'industrie de la distribution ont progressé plus fortement que les prix agricoles, entraînant une inflation supplémentaire injustifiée pour les consommateurs. Le consommateur est lui aussi lésé. En un an, les prix des produits alimentaires ont bondi de 2 %, soit leur plus forte hausse depuis 2012. Cette augmentation atteint 5,2 % pour les produits frais, et jusqu'à 10 % même pour certains autres produits. Nous l'avions dénoncé lors des débats sur le projet de loi Égalim. De simples engagements volontaires à mettre en oeuvre des chartes et des plans, ou encore des indicateurs ne peuvent remplacer de véritables outils contraignants de régulation des marchés agricoles. D'autant qu'aujourd'hui ces centrales organisent leur extraterritorialité, à l'image d'un groupe français qui a pour slogan « vous savez que vous achetez moins cher » et qui, pour ce faire, développe à partir de Bruxelles, une centrale d'achat qui négocie ouvertement les prix pour le marché français. De la sorte, il devient possible de s'affranchir de certaines règles françaises : droit de la concurrence, délais de paiement ... Ce groupe a terminé l'année 2018 avec un chiffre d'affaires de 37,75 milliards d'euros, en progression de 1,5 % par rapport à l'année précédente. Enfin, certains mécanismes, comme le relèvement du seuil de revente à perte et l'encadrement des promotions, ont eu des effets contraires à ceux qui sont recherchés, cela a déjà été dit. Ainsi, les sénateurs, mais aussi les associations de consommateurs, comme l'UFC-Que Choisir, ou encore les organisations syndicales agricoles telles que la Confédération paysanne et la FNSEA s'accordent pour dire que ces outils n'ont pas fonctionné, voire qu'ils ont eu des effets néfastes sur l'emploi des PME. Pour l'UFC-Que Choisir et la Confédération paysanne, le système du seuil de revente à perte est un « chèque en blanc de 1,6 milliard d'euros à la grande distribution » sur deux ans et un « chèque en bois pour les agriculteurs ». La hausse du seuil de revente à perte a modifié la composition des linéaires selon les types de marque dans les grandes surfaces et a eu pour effet de revaloriser les produits des grandes marques et sous marques de distributeurs dans les rayons au détriment des produits des PME de l'industrie agroalimentaire. Les ventes en valeur des produits des PME ont diminué de 3,7 points entre 2018 et 2019, tandis que pour les produits sous marques de distributeurs, la croissance de ces ventes a enregistré une augmentation de 0,3 point. Concernant l'encadrement des promotions, il y a eu purement et simplement un détournement du dispositif le développement de nouvelles offres commerciales. Il en est ainsi de ce qui est maintenant communément appelé le « cagnottage », technique de fidélisation qui consiste pour les distributeurs à proposer l'achat de certains produits et des réductions, dont le montant peut être reporté sur une carte. Il également du déplacement de la promotion : l'encadrement ne s'appliquant que sur un même produit, la grande distribution a simplement déplacé son offre sur des produits annexes. Si les produits sont différents, de fait, l'encadrement ne s'applique pas. Face à ce constat, la proposition de loi, signée par l'ensemble des membres de la commission des affaires économiques, a le mérite de répondre dans l'urgence aux défaillances les plus criantes de la loi Égalim. Ses dispositions sont d'application directe

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, issue des États généraux de l'alimentation, la loi Égalim a suscité de grands espoirs. Un an après le début de son application et au milieu de l'expérimentation prévue, force est de constater qu'elle peine encore à porter ses fruits, et des effets pervers sont apparus. La présente proposition de loi résultant des travaux du groupe de suivi de la loi Égalim tend à corriger ces derniers. Elle comporte trois mesures d'urgence : la fin de l'encadrement des promotions dans certains cas, notamment pour des produits saisonniers marqués, l'expérimentation d'une clause de révision automatique des prix, et une disposition concernant le droit coopératif. Je souhaite m'attarder sur la deuxième mesure, l'expérimentation de la conclusion d'une clause de révision automatique des prix. En effet, le mécanisme actuel de révision des prix paraît trop lourd pour que les acteurs s'en emparent. Librement consentie par les parties, cette clause fonctionnera à la hausse comme à la baisse au cours de l'année. La nécessité d'un tel mécanisme est parfaitement illustrée par la forte augmentation du prix du porc, conséquence de la peste porcine africaine qui décime actuellement les élevages chinois. En 2019, le prix du porc a augmenté de près de 50 %. De tels à-coups sont susceptibles de mettre en péril l'équilibre de certains contrats et la pérennité des entreprises, en particulier des PME. C'est notamment le cas des producteurs de charcuterie qui achètent le porc au prix du marché, mais revendent leurs produits à un prix fixé par un contrat qu'ils ont conclu antérieurement avec le distributeur. La situation devient ainsi intenable pour bon nombre d'entre eux. La clause de révision automatique des prix nous semble être de nature à permettre aux contrats de rester en phase avec les réalités du marché et à garantir plus de justice. En outre, nous saluons la proposition de suppression de la disposition prévoyant la possibilité d'engager la responsabilité des coopératives pour les rémunérations abusivement basses des apports. Cette transposition du code de commerce vers le code rural de la notion de prix abusivement bas nous paraît, d'une part, dépasser le cadre de l'habilitation législative conférée au Gouvernement, d'autre part, être parfaitement inadaptée au système coopératif. Le groupe Les Indépendants soutient et votera cette proposition de loi, qui illustre parfaitement le travail de la Haute Assemblée. Le groupe de suivi de la loi Égalim est animé par la seule volonté

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la loi Égalim est l'aboutissement de longs mois de discussions. Elle porte en elle l'espoir de lendemains meilleurs pour des producteurs français en grande détresse. Aussi, dès sa promulgation, fin octobre 2018, le Sénat a souhaité mettre en place un groupe de suivi. J'ai eu le plaisir de participer, avec mes collègues Daniel Gremillet et Michel Raison, à ces rencontres régulières avec les acteurs économiques. Au cours de ces entretiens, ces fameux « effets de bord » préjudiciables aux entreprises sont apparus. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise à les corriger sans attendre, mais sans pour autant préjuger l'efficacité globale de la loi qui ne pourra être appréhendée qu'à l'issue de la période expérimentale, dans un an. Les préconisations d'étape sont de trois ordres : l'encadrement des promotions, la clause de révision des prix et le cadre de l'ordonnance sur les coopératives. Dès le début 2019, la grande distribution, pourtant bénéficiaire de la hausse du SRP, a choisi de baisser les prix sur les produits sous marques de distributeurs, ainsi que sur ceux des rayons non alimentaires, engageant ainsi une nouvelle guerre des prix entre distributeurs. Quant aux mesures d'encadrement des promotions, elles ont été rapidement contournées, en jouant sur les cagnottes des cartes fidélité et en associant des produits différents. La grande distribution a ainsi cherché à se reconstituer des marges. À ce stade de la mise en oeuvre de la loi, vous-même, monsieur le ministre, vous constatez que le compte n'y est pas. Le fameux relèvement du seuil de revente à perte qui devait donner de nouvelles marges aux industriels pour mieux rémunérer les producteurs, selon la théorie du ruissellement, ne se vérifie pas. Où sont donc passés les bénéfices de l'inflation et du SRP, pourtant bel et bien payés par les consommateurs ? L'un des grands gagnants de la loi, à ce stade, c'est peut-être aussi l'État, grâce aux recettes supplémentaires de TVA liées au relèvement du SRP. SRP. Le paradoxe de la loi Égalim, que nous souhaitons corriger aujourd'hui, c'est qu'elle pénalise, au final, les entreprises les plus proches des agriculteurs. Ce sont désormais les grandes marques et les MDD qui sont privilégiées dans les linéaires des grandes surfaces. Les PME alimentaires ne sont plus au coeur de la stratégie des distributeurs. Elles se trouvent reléguées, et leur croissance a brutalement ralenti depuis le début d'année. En encadrant plus strictement toute promotion, la loi a introduit un biais anticoncurrentiel à leur détriment : elles ne peuvent pas rivaliser avec les budgets marketing des grandes marques. À défaut de diffuser un spot publicitaire à la télévision, elles faisaient, jusqu'alors, des promotions en magasin. La loi les a en partie privées de cet outil. Certaines ont ainsi perdu jusqu'à 50 % de leur chiffre d'affaires depuis le début de l'année dernière. Pour remédier à ces difficultés, de loi vise à sortir les produits saisonniers de l'encadrement en volume des promotions, de manière à permettre de mieux écouler les stocks.

revenir à un modèle dans lequel les coopératives agricoles ne sont pas assimilées à des entreprises privées, conformément à la volonté du législateur exprimée dans le cadre du vote des ordonnances. Monsieur le ministre, l'urgence est bien réelle pour la survie de ces entreprises. Pour ces motifs, le groupe Union Centriste soutiendra cette proposition en souhaitant que les travaux du groupe de suivi ne s'arrêtent pas là et qu'ils reviennent sur les questions du revenu agricole, de la compétitivité des entreprises, du surcroît des charges imposées, la restauration collective et peut-être et surtout sur le respect de l'article 44, mesure clé de voûte face à la concurrence déloyale de produits qui ne respecte pas les exigences européennes de production et exerce une pression à la baisse sur l'ensemble des produits agricoles en France. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à mon tour de féliciter le travail mené depuis l'adoption de la loi par Daniel Gremillet, Michel Raison, Anne-Catherine Loisier, mais aussi tous les membres du groupe de suivi de la commission des affaires économiques. Ce travail de

à examiner. Nous sommes plus que jamais dans notre rôle institutionnel de contrôle du Gouvernement qui aboutit, si besoin est, à des propositions de modification de cette loi. Cette action sénatoriale se manifeste aussi, monsieur le ministre, dans le strict respect du champ de l'ordonnance. Le recours accru aux ordonnances opère un dessaisissement inquiétant du Parlement. Mes chers collègues,

entrent en application sans ratification et les instruments de contrôle du Parlement sont limités, y compris si le Gouvernement sort du champ de son habilitation. Ainsi, rappeler au Gouvernement qu'il doit strictement se limiter au champ de l'habilitation qui lui a été accordée par le Parlement au moment de l'adoption de la loi, comme le fait cette proposition de loi, c'est aussi exercer un travail de contrôle parlementaire nécessaire. Venons-en au bilan de la loi Égalim à ce stade. Vous le savez, monsieur le ministre, le Sénat a émis très tôt des doutes sur l'efficacité de cette loi, notamment sur le SRP et sur cette fameuse cascade. Mais non, nous n'avons pas voulu détricoter, dans cette proposition de loi, l'ensemble de la loi de la loi qui a été adoptée ! En effet, nous voulons, comme vous, aller jusqu'au bout de l'expérimentation et nous voulons prendre le temps, chère Noëlle Rauscent, de mesurer les effets réels de la loi. Nos auditions et nos déplacements nous ont permis de rencontrer les acteurs de terrain. Ce sont eux Ce sont eux les mieux placés pour juger de l'efficacité de la loi. Certaines entreprises accusent des reculs considérables de leur chiffre d'affaires compte tenu de l'encadrement des promotions

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en juillet 2018, je disais ici, au nom de mon groupe, notre scepticisme quant aux effets réels que pouvait avoir la loi Égalim sur la modification de la répartition de la valeur créée tout au long de la chaîne, qui va du producteur au distributeur. Je salue l'initiative de la présidente de la commission des affaires économiques qui a, sans tarder, engagé une évaluation des premiers effets de ce texte à partir du round de négociations commerciales 2018-2019. Je suis un fervent promoteur des démarches d'évaluation des politiques publiques et le Sénat donne en l'espèce l'exemple, en lien très fort avec les territoires et leurs acteurs, d'une évaluation de l'efficacité du travail législatif et gouvernemental. étaient une belle promesse à laquelle nous avons voulu croire ! Mais pour ce qui est des prix et des revenus, ils sont venus se fracasser sur la réalité d'un contexte économique tendu qui a conduit à une baisse globale constatée des prix de l'ordre de 0,4 % selon l'Observatoire de la formation des prix et des marges. Les transformateurs ne s'y retrouvent pas et les producteurs, sauf exception tenant plus de la conjoncture internationale que des effets de cette loi, n'ont pas vu l'amorce d'une amélioration de leur revenu. Dès lors, et même si nous n'en sommes qu'au mitan de la période d'expérimentation, il était sain et responsable de réagir, afin de corriger certains mécanismes, de toute évidence dévoyés par la pratique, bien éloignés de l'esprit du législateur de la

de la bouche d'un représentant de la filière « gras-volailles festives » : le seuil de revente à perte a été très préjudiciable pour les productions saisonnières. Il a donné lieu à des contournements inacceptables que vos services doivent repérer et sanctionner. Je sais que vous vous y employez. Le SRP s'est aussi traduit négativement pour certains vins dont l'acte d'achat est étroitement lié aux périodes de fêtes. Le président d'une grande coopérative viticole gersoise vous l'a aussi dit. Il faudra que la liste des produits dérogatoires au SRP prévue par le texte que nous allons voter aujourd'hui tienne compte des pratiques saisonnières des consommateurs dans leur ensemble. Les professionnels et leurs représentants devront être étroitement associés à ce travail de définition. Aux grandes difficultés éprouvées par la filière « gras » depuis 2015- notamment les deux épisodes catastrophiques de grippe aviaire -ne doivent pas s'ajouter les effets délétères du SRP.

Pour dire les choses plus prosaïquement, les agriculteurs ne doivent pas payer pour la guerre menée dans la filière aéronautique. Ce texte prévoit ensuite de conduire une expérimentation en adaptant les mécanismes de la clause de révision des prix des contrats de plus de trois mois passés entre distributeurs et entreprises ciblage des produits finis composés à plus de 50 % d'un produit agricole, plus grande réactivité et automaticité de la révision à la hausse ou à la baisse, simplification de la procédure ont présidé à l'introduction de l'article 2. L'expérimentation durera trois ans et les produits seront arrêtés par décret. Tout en étant favorables à cette expérimentation, nous pensons que le risque est grand de voir le rapport de force continuer de prévaloir, les seuils de déclenchement étant renvoyés à la négociation entre les parties. Enfin, il nous paraissait nécessaire, nonobstant les questions de fond relatives à la nature même du contrat liant le coopérateur à sa coopérative agricole, que le champ de l'habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance, fixé par le législateur, soit strictement Pour terminer, je me réjouis que ce texte, qui concerne la vie de nos territoires, ait réuni des signataires de tous les groupes politiques de la Haute Assemblée, sans exception. J'espère que le Gouvernement voudra le faire prospérer à l'Assemblée nationale, dans l'intérêt des entreprises et des exploitations concernées. loi laisse entière la question du revenu des agriculteurs à laquelle le Gouvernement, notamment à travers la PAC, devra apporter des réponses à la hauteur des enjeux et de la situation difficile que vivent nombre d'entre eux.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier la commission des affaires économiques de la création du groupe de suivi de la loi Égalim auquel j'appartiens,

Sur le terrain, les maires nous rappellent d'autres exemples, comme le fiasco de la réforme des rythmes scolaires et la limitation de la vitesse à 80 kilomètres par heure. Comment leur répondre ? Comment leur expliquer que, trop souvent, les textes s'enchaînent et que l'énorme travail réalisé en commission est quelquefois balayé d'un revers de main pour des raisons d'entêtement politique ?

Grâce à des réunions thématisées, les enjeux ont été posés et chacun a pu s'exprimer. Jusque-là, tout allait bien : il s'agissait d'une posture innovante, à la hauteur des défis de notre agriculture. Malheureusement, les bonnes intentions se sont arrêtées là. Dès l'examen du projet de loi, comme très souvent, nous avons assisté à un véritable déni de démocratie. Le Sénat vous avait averti des conséquences de certaines mesures, car nous sommes proches des territoires et de leurs acteurs. Les responsables professionnels, qui ont aussi adopté une posture constructive en s'investissant dans les États généraux, nous avaient alertés sur certains points d'achoppement. Nous avons relayé ces craintes, mais nous n'avons pas été Premier écueil : pourquoi généraliser une mesure destinée à gérer une problématique particulière, à savoir la commercialisation de certains produits trop conditionnés à des ventes en promotion ? Pour répondre à ce contexte de menace pour nos éleveurs, par exemple dans la filière porcine, la loi a généralisé la limitation des ventes sous promotion sans tenir compte d'un argument soulevé durant les auditions

les petites entreprises, souvent familiales, qui ne peuvent se payer de publicité et qui vivaient grâce au système des promotions, sont en grand danger. raison pour laquelle nous demandons unanimement que seule l'autorité compétente, à savoir la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, définisse le caractère saisonnier. Faisons confiance à nos administrations, si toutefois elles sont libres de se prononcer.

Cela nous oblige à réfléchir et à revenir sur un sujet de fond : l'avenir de notre agriculture. Voulons-nous maintenir les structures familiales ou privilégier les grosses unités ?

Vous l'avez compris, la loi Égalim, fruit d'une excellente méthode, s'est arrêtée en marche. Notre posture n'est pas politicienne. Seul l'avenir de notre agriculture compte.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, persuadé que l'agriculture et l'alimentation sont l'affaire de tous, le groupe Les Indépendants s'était mobilisé tout au long de l'examen de la loi Égalim pour défendre un modèle agricole économiquement viable et écologiquement responsable. L'agriculture est au coeur de la société française, tant par son importance économique que par le profond attachement de nos concitoyens à son égard. Il s'agit cependant d'un secteur qui connaît de fortes mutations et dans lequel la souffrance perdure.

La logique promotionnelle contient le risque d'une rémunération au rabais. Pour en sortir, la loi Égalim prévoit un strict encadrement des promotions, notamment leur limitation en volume. L'objectif est louable, mais il a un effet dévastateur sur les produits saisonniers dont la promotion représente une part essentielle des ventes. Des produits comme le foie gras ou le lapin ne sont achetés qu'à certaines périodes. Hors celles-ci, seules les promotions sont à même de susciter l'achat. La mesure d'encadrement ne convient donc pas aux secteurs à saisonnalité marquée. Les différentes auditions laissent penser que d'autres ajustements de la loi Égalim pourraient s'avérer nécessaires. Les mesures contenues dans cette proposition de loi, ainsi que leur caractère limité, démontrent non seulement l'attention que porte le Sénat au monde agricole, mais aussi son écoute et son esprit constructif. Je souhaite féliciter Daniel Gremillet, Michel Raison et Anne-Catherine Loisier pour leur action déterminée. Le groupe Les Indépendants soutient les objectifs de cette proposition de loi. L'agriculture est l'un des atouts les plus précieux de notre pays ; nous souhaitons le voir prospérer et nous y travaillerons.

en septembre 2018, à cette même tribune, j'avais estimé que le projet de loi Égalim était décevant sur le fond, car il n'était pas l'expression des conclusions des États généraux de l'alimentation. Il détricotait ce qui fonctionne, comme la sécurisation des pratiques contractuelles et des engagements pluriannuels adaptés à la filière viticole. Je l'avais jugé décevant aussi sur la forme : la CMP n'a pas été conclusive, car la majorité de l'Assemblée nationale est restée figée sur les positions du Gouvernement, en contradiction parfois avec ses propres votes. Les sénateurs ne pouvaient accepter que leur travail soit balayé d'un revers de main par les députés, alors que leur regard initial était constructif et bienveillant. était décevant, voire alarmant, pour l'économie. Ce rendez-vous devait être le moment de revaloriser le revenu de nos agriculteurs qui souffrent encore trop. Il devait permettre d'inverser le rapport de force entre les producteurs et la grande distribution.

Ainsi, la commission des affaires économiques a adopté, le 30 octobre dernier, le rapport d'information n° 89 du groupe de suivi de la loi Égalim. Malheureusement, comme son titre l'indique, un an après, le compte n'y est pas. Sur ce point au moins, monsieur le ministre, nous sommes d'accord. La proposition de loi que nous étudions aujourd'hui, et que j'ai bien évidemment cosignée, tire les conclusions du premier bilan de cette loi réalisé par la commission des affaires économiques, sous la direction de Michel Raison et Anne-Catherine Loisier que je félicite pour leurs travaux et leur implication. Trois effets particulièrement problématiques, notamment pour les PME, ont été soulevés : tout d'abord, certaines d'entre elles accusent un recul considérable de leur activité compte tenu de l'encadrement des promotions en volume- 25 % de leur chiffre d'affaires prévisionnel certains industriels peinent à renégocier leurs contrats avec leurs distributeurs en cours d'année en cas de hausse des cours des matières premières agricoles entrant dans la composition de leurs produits

Il est aujourd'hui un peu tôt pour dresser un bilan exhaustif et incontestable de la loi Égalim, même si des doutes demeurent. Ainsi, le groupe de suivi poursuivra ses travaux de contrôle en 2020. Toutefois, son premier rapport est clair : des PME et des ETI sont très fragilisées par la loi. Au bout de la chaîne, ce sont bien les producteurs agricoles qui verront leurs revenus pâtir de la baisse d'activité de ces entreprises. Si les failles sont d'ores et déjà repérées, pourquoi ne pas agir tout de suite ? Tout le monde souhaite que les agriculteurs soient mieux rémunérés à court terme. Cette proposition de loi entend justement renforcer ses chances de succès en limitant ses effets de bord et en proposant une amélioration. La commission a appuyé cette démarche. Je soutiens les mesures de cette proposition de loi et le groupe Union Centriste votera en faveur de ce texte. La parole

pour un transfert de ces bénéfices sur les produits agricoles, l'encadrement des promotions à 25 % pour tout produit en valeur et en volume et le report des augmentations des matières premières sur les prix finaux dans les grands magasins.

Certaines mesures déstabilisent très clairement les PME et les ETI des territoires et n'apportent pas de marge supplémentaire à nos agriculteurs. La revalorisation du SRP de 10 % qui visait à renforcer l'équilibre général des négociations au profit des entreprises et des agriculteurs et à augmenter les prix et les revenus complémentaires des agriculteurs a été un échec. penser que la grande distribution, qui possède 92 % de parts de marché, allait transférer des marges supplémentaires des SRP pour augmenter le prix d'achat des produits agricoles ou des TPE était illusoire.

final, ces sociétés se sont retrouvées en difficulté, ce qui est absolument anormal. De plus, on s'aperçoit que les promotions pratiquées par les TPE ou par les entreprises familiales de nos territoires sont un moyen de publicité efficace, sans doute l'un des seuls dont elles disposent.

Devant l'urgence et la détresse des entreprises familiales de nos territoires qui ont vu leur chiffre d'affaires et leur bénéfice fondre, le groupe de suivi a vite réagi. Je tiens à l'en féliciter.

l'expérimentation d'une clause automatique de révision des prix tous les trois mois, en fonction des cours ; la suppression de la possibilité pour les juges de sanctionner financièrement des coopératives ayant pratiqué une politique de prix extrêmement basse. Il est indispensable de maintenir et de développer le tissu de PME sur les territoires qui paient de la TVA, des impôts et des charges sociales. Ce sont elles qui génèrent de l'emploi sur les territoires et créent la richesse du pays.

années. Les industriels ont toujours eu une logique de préservation des marges pour leurs fournisseurs, permettant d'assurer de la stabilité et de la continuité. Or la grande distribution n'a jamais partagé cette philosophie. Il faut que cette mécanique change. change. L'agriculture française doit aussi se réformer et s'adapter aux évolutions et aux besoins du consommateur. Nous en sommes bien conscients. Cette proposition de loi vient corriger certains errements de la loi Égalim. J'ai bien entendu, monsieur le ministre, que le Gouvernement y était défavorable. J'espère simplement que vous reverrez votre position ou que vous nous proposerez d'autres solutions. Nous ne pouvons en rester à la situation actuelle. Je voterai cette proposition

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il est rare qu'une proposition de loi reflète une position partagée quasi unanimement sur les travées de notre hémicycle. je tiens à remercier Daniel Gremillet de nous avoir associés à ce texte totalement transpartisan, cosigné par une centaine de collègues, issus de tous les groupes. Lorsque les clivages traditionnels entre nos groupes sont ainsi surmontés, c'est que l'enjeu est suffisamment fort pour nous inviter à faire cause commune. Et lorsque notre assemblée est ainsi homogène dans son expression, il serait bon que le Gouvernement l'entende. Le constat d'échec de la loi Égalim que nous faisons tous aujourd'hui n'est malheureusement pas une surprise. Si les États généraux de l'alimentation avaient suscité de vrais espoirs, le texte censé les traduire s'est avéré des plus décevants, sur les volets tant des revenus des agriculteurs que de l'alimentation. Très vite, il nous a semblé nécessaire de constituer, au sein de la commission des affaires économiques, un groupe de suivi de cette loi, afin d'en analyser la portée réelle. Les travaux de ce groupe ont permis de mettre en évidence les effets néfastes de ce texte qui ont affecté encore davantage les agriculteurs, plus particulièrement les PME, grandes victimes de la loi Égalim. Ainsi, le relèvement du seuil de revente à perte de 10 % sur les produits alimentaires et l'encadrement des promotions n'auront pas permis d'augmenter le revenu des agriculteurs. Le prix d'achat aux fournisseurs en 2019 aura même diminué de 0,4 % selon l'Observatoire de la formation des prix et des marges. En conclusion, les auteurs du rapport de suivi ont souligné que « la loi Égalim aura l'effet paradoxal de pénaliser les acteurs les plus proches des agriculteurs français et qui, souvent, sont les plus créateurs d'emplois ». Il était donc indispensable de légiférer de nouveau pour corriger sans attendre les effets les plus négatifs de ce texte. Cette proposition de loi transcrit les préconisations du groupe de suivi. Trois problèmes doivent doivent être « résolus avec urgence » pour ne pas mettre en difficulté les entreprises françaises de l'agroalimentaire et les producteurs agricoles : les difficultés majeures posées par l'encadrement des promotions pour les PME ; les effets de la clause de renégociation des prix jugés non satisfaisants ; la réforme considérée par certains comme trop extensive en matière de droit des coopératives agricoles sur la base de l'habilitation par ordonnance prévue dans la loi Égalim. Ces problématiques se traduisent très directement dans les trois articles de la proposition de loi.

qui permet d'ajuster mécaniquement le prix d'achat contractuel à la hausse comme à la baisse. C'est le cas du porc, dont le cours a augmenté de 45 % entre janvier et octobre 2019, alors même que le coût de la matière première constitue 70 % du coût de revient de l'industrie charcutière, ou encore des pâtes alimentaires, affectées par une augmentation du cours mondial du blé dur de 25 % en six mois. Si le travail en commission a eu le mérite de simplifier le dispositif retenu, l'une des modifications opérées par rapport au texte initial risque d'avoir des effets non désirés : en renvoyant les seuils de déclenchement de la clause à la négociation entre les parties, elle pose une fois de plus la question du rapport de force lors de tels échanges. La grande distribution risque d'être intraitable sur ses seuils, rendant leur activation sûrement difficile, sinon très encadrée. L'article 3 tend à la suppression du régime des prix abusivement bas. À cet endroit du texte, j'aurai une approche légèrement différente de celle de mes collègues. Je les rejoins sur le fait que le Gouvernement est allé au-delà du champ de l'habilitation que lui donnait l'article 11 de la en modifiant le code rural, alors que la loi ne citait que le code du commerce. Comme eux, je suis attaché aux droits du Parlement. Trop souvent, ces dernières années, nous avons contesté la confiscation des débats parlementaires par le recours aux ordonnances. Je suis également très attaché au modèle coopératif et je conçois que mes collègues soient choqués par l'assimilation, de fait, des coopératives à des sociétés commerciales. Toutefois, les dispositions supprimées par l'article 3 permettraient à des associés coopérateurs se sentant lésés du fait d'une rémunération abusivement basse de leurs apports au regard des indicateurs agricoles de pouvoir mettre fin à cette situation ou d'obtenir réparation en justice. Elles constitueraient donc une parade contre certaines pratiques affectant le revenu des agriculteurs. Ces derniers, nous le savons, se sentent parfois impuissants, notamment lorsqu'ils appartiennent à de très grosses coopératives s'apparentant à des géants de l'agroalimentaire. Il ne s'agit pas de remettre en cause l'esprit coopératif, car le dispositif, tel qu'il est prévu dans la loi, reste relativement lourd et ne s'appliquerait donc que dans certains cas extrêmes. En effet, l'action en justice doit être introduite par le ministre de l'économie, après l'avis motivé du ministre de l'agriculture et du Haut Conseil

dans ces situations. Toutefois, dans un souci de maintenir cette belle unanimité sur ce texte et me retrouvant, à cette nuance près, complètement dans la démarche des auteurs de cette proposition de loi, j'ai retiré mon amendement visant à supprimer l'alinéa 2 de l'article 3. Mes chers collègues, la loi Égalim, malgré tout le travail effectué en amont, notamment au travers des États généraux, est en échec sur ses principaux objectifs. Il nous appartient aujourd'hui, à travers cette proposition de loi, d'en corriger les effets les plus néfastes. Les membres du groupe socialiste et républicain voteront cette proposition de loi transpartisane.

comme nombre d'entre nous, je suis élue d'un département où l'agriculture est un moteur essentiel de la vie économique : 7,5 % de la population active travaille dans ce secteur, générant un chiffre d'affaires de 720 millions d'euros, d'euros, comparable à celui de l'industrie agroalimentaire. Au-delà de son poids économique, nous avons un attachement viscéral à cette activité si particulière qui façonne notre territoire et dont il ne faut pas oublier l'objectif essentiel produire, nourrir, et pouvoir vivre de son travail. La loi Égalim est un rendez-vous manqué pour les agriculteurs. Elle aborde les enjeux liés à l'alimentation, aux relations commerciales entre les producteurs et les distributeurs de manière imparfaite. Les réponses apportées à leur précarisation ne sont pas à la hauteur, la loi n'ayant un effet que sur un cinquième des recettes des agriculteurs et quelques filières. Aussi, je veux saluer la qualité des travaux du groupe de suivi, qui nous conduit à débattre cet après-midi de cette proposition de loi, largement cosignée. Elle est attendue par le monde agricole, dont de nombreuses PME et entreprises de taille intermédiaire. En effet, certaines conséquences négatives de la loi Égalim sont déjà clairement identifiées. C'est le cas notamment du recul de l'activité lié à l'encadrement des promotions en volume, dont les effets sont particulièrement douloureux pour les produits à forte saisonnalité, avec des baisses de chiffre d'affaires allant jusqu'à 50 % et au-delà. Comme le souligne Daniel Gremillet, auteur de la proposition de loi, « sans soutien promotionnel, les ventes s'effondrent. » Allons-nous laisser s'affaiblir puis disparaître ces productions ? De plus, les difficultés persistent dans les mécanismes de renégociation des prix et des contrats en cours d'année. Il est significatif que les industriels porcins aient préféré ne pas y recourir l'an passé, en raison de leur lourdeur et de leur faible protection. Monsieur le ministre, vous avez là, clé en main, des solutions aux « effets de bord » que relève M. le rapporteur, Michel Raison. Vous le savez, le monde agricole est en crise. Nous le répétons sans honte et le répéterons sans relâche, le monde agricole est en crise depuis trop longtemps.

le développement de l'agri-bashing conduisent les jeunes générations à faire le choix rationnel de ne pas se lancer dans cette voie. L'enjeu du renouvellement des générations n'a jamais été aussi important : un tiers des agriculteurs a plus de 50 ans. ans. Notre pays est déjà devenu la troisième puissance agricole, derrière l'Allemagne et les Pays-Bas. Faudra-t-il attendre sans bouger que notre excédent commercial agricole disparaisse du fait de la concurrence européenne ? Quels signaux supplémentaires faut-il pour réveiller les consciences et agir ? Évidemment, l'amélioration de la condition des agriculteurs ne se fera pas du jour au lendemain. Les changements proposés doivent être apportés progressivement et corrigés au fur et à mesure lorsqu'ils produisent des effets négatifs. Le bon sens fait les hommes capables » disait Napoléon. Du bon sens, les agriculteurs en ont ! Il est temps que notre pays retrouve la fierté de son agriculture. Aussi, monsieur le ministre, je vous invite à vous appuyer sur la vigilance du Sénat

pour demander des dérogations. Nous serons ravis qu'elles puissent être sauvées dans nos territoires.

pieds sur terre. En effet, nous voilà réunis pour remettre dans la loi ce que nous y avions déjà inscrit en première et unique lecture, mais qui fut retoqué. Il s'agit d'éviter le mécanisme d'habilitation à légiférer par ordonnances, qui a empêché le débat, ce que le monde agricole paye maintenant fort cher. S'agissant du seuil de revente à perte et de l'encadrement des promotions, ces mesures phares de l'article 15 entrées en vigueur le 12 décembre 2018 n'ont pas donné les effets escomptés, bien au contraire. L'Assemblée nationale, dans son rapport d'information du 29 mai dernier sur l'application de la loi Égalim, a rappelé un courrier du 12 février 2019 cosigné par les industriels et les agriculteurs, considéraient que l'absence d'encadrement par l'ordonnance des annonces non chiffrées de promotion, telles les formules « prix-choc » ou « prix bas » et les propositions de cagnottage portant sur l'ensemble d'un rayon limitaient significativement les effets de l'ordonnance. Et les rapporteurs de rappeler alors : le dispositif « était prévu pour une durée de deux ans : à l'issue de ce délai et après en avoir analysé les effets, il sera toujours temps de l'aménager, de le supprimer ou de le pérenniser. » Mais ce temps-là est trop long, au vu des dysfonctionnements, qui sont apparus très vite, mettant en péril nos PME de l'agroalimentaire et, donc, nos agriculteurs. Telles sont les raisons pour lesquelles les